et Républicain. Oui, la situation sanitaire est grave. Oui, des dispositions contraignantes devaient être prises, comme dans tous les pays européens. Oui, il faut freiner la circulation du virus pour permettre aux soignants de tenir. Oui, nous devons faire preuve de responsabilité, comme nous l'avons fait en votant la déclaration du Gouvernement. Toutefois, encore faut-il que les décisions soient logiques et équitables ! Comment justifier la fermeture des petits commerces, qui appliquent les protocoles sanitaires, au prétexte qu'ils ne seraient pas « essentiels » ? Comment justifier qu'acheter un fer à repasser dans une grande enseigne soit plus « essentiel » qu'acheter un livre en librairie ? Comment justifier que monter dans un bus pour aller travailler soit plus sûr que faire une balade en forêt à plus d'un kilomètre de chez soi ? Aussi, ma question est simple : où est la logique ? Quelle en est l'efficacité ?

L'important n'est pas de comprendre les frustrations des uns et des autres ; c'est que les décisions soient acceptées. Or, pour qu'elles soient acceptables, il faut qu'elles soient compréhensibles. Et si cette acceptabilité passait par un changement de méthode ? Voici quelques propositions : changer la logique en privilégiant les protocoles sanitaires, plutôt qu'en raisonnant par « produits essentiels » ou par type de commerce

d'aller d'état d'urgence en état d'urgence sans concertation, modifiez la gouvernance de cette crise en vous appuyant sur le Parlement, plutôt qu'en lui donnant la leçon, comme hier soir, à l'Assemblée nationale.

Pour que la responsabilité soit partagée, encore faut-il que la décision le soit aussi. La parole

Monsieur le ministre de l'économie, la deuxième vague de l'épidémie de covid-19 frappe notre pays de plein fouet. Le nombre des personnes infectées dépasse les chiffres du mois de mars dernier, et les indicateurs sont au rouge. Face à la gravité de la situation, le Gouvernement a décidé par décret, le 29 octobre dernier, et selon des critères bien flous, de fermer les commerces dits « non essentiels », parmi lesquels nombre de petits commerces de proximité. Cette décision soulève une incompréhension doublée d'un sentiment d'injustice pour des professionnels qui avaient mis en place des mesures garantissant la sécurité sanitaire de leurs salariés et de leurs clients : flacons de gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire, nombre limité de clients dans les locaux Je redoute que cette fermeture ne représente le coup de grâce pour l'économie locale. Alors que les mastodontes du commerce en ligne et de la grande distribution restent ouverts, cette différence de traitement introduit une discrimination.

Il lui serait possible d'accueillir un client à la fois en appliquant des règles sanitaires strictes, sans pour autant contribuer à propager le virus. Ailleurs, des maires ont pris, en toute illégalité, des arrêtés pour rouvrir ces commerces, que l'Association des maires de France demande, dans un communiqué, le réexamen de la notion de commerce de première nécessité. Pour répondre à la grogne, vous avez annoncé dimanche un fonds de 100 millions d'euros d'aides pour accélérer la digitalisation et mettre en place un service de, accompagné d'incitations financières. Afin de leur donner une chance de survivre à ce nouveau confinement, et parce qu'ils assurent un service indispensable à la vie sociale et économique de nos communes et de nos territoires, le groupe RDSE et moi-même vous demandons, monsieur le ministre, d'autoriser l'ouverture des petits commerces de proximité par dérogation accordée par le préfet, à la demande des maires. La mise en place de ce système dérogatoire remettra au coeur du dispositif le couple maire-préfet.

Le confinement est devenu indispensable pour la sécurité sanitaire, mais les petits commerçants payent un lourd tribut. Pour la seconde fois, ils sont obligés de fermer boutique et vivent une situation dramatique. De plus, les mesures mises en place introduisent une inégalité de traitement avec les grandes et moyennes surfaces, d'une part, et avec les géants du numérique, d'autre part. C'est une inégalité insoutenable. Comment accepter cette situation invraisemblable : nos petits commerces sont obligés de fermer, et, en parallèle, des entrepôts d'Amazon s'implantent un peu partout sur notre territoire ? Ce modèle économique n'est pas durable. Il est à l'origine de dizaines de milliers de destructions d'emplois dans les commerces traditionnels.

Demander la relocalisation de nos productions et appeler à plus de souveraineté, c'est bien. Mais il ne faut pas pleurer la mort des petits commerces de proximité et, en parallèle, autoriser des implantations et des extensions de grandes surfaces et accepter la construction de vingt nouveaux entrepôts géants d'Amazon un peu partout en France relève bien de la responsabilité des élus locaux d'accepter, ou non, l'implantation de ces sites sur leur commune. C'est le cas à Belin-Béliet, en Gironde, où le géant chinois Alibaba va implanter 71 000 mètres carrés d'entrepôts logistiques en plein parc naturel régional, mais aussi à Ensisheim, dans le Haut-Rhin, ou encore à Montbert, en Loire Atlantique. La liste est longue ! Je pourrais également parler des conditions sanitaires des salariés dans la vente en ligne. Monsieur le ministre, pour enfin trouver le chemin d'un modèle économique juste et résilient, soyons efficaces sans attendre. À quand un gel des implantations d'entrepôts de vente en ligne, comme le demande la Convention citoyenne pour le climat, et un moratoire sur leurs ouvertures ? Oui, à quand ? À quand une contribution exceptionnelle d'Amazon et des grandes surfaces en faveur des commerçants et artisans obligés de fermer ? je vous remercie

reconfinement, que nous pouvons qualifier de partiel. Les écoles, les collèges et les lycées sont ouverts ; certains commerces, les grandes surfaces, les GAFA et les grands groupes qui livrent les foyers travaillent, tandis que d'autres sont fermés.

Si vous mettez le doigt là-dedans, vous n'en sortirez jamais ! Tous les jours apparaîtront de nouveaux produits de première nécessité, forts d'arguments tenant la route. La boussole, ce doit être la sécurité sanitaire.

suscitent légitimement. Hier encore, plus de 430 personnes sont mortes en France. Cette maladie touche toutes les tranches d'âge,

est à Mme Dominique Estrosi Sassone, pour le groupe Les Républicains. Dites à mes enfants que je les aime » : tels sont les derniers mots prononcés par Simone, lâchement assassinée, comme Nadine et Vincent, en plein coeur de la basilique Notre-Dame de Nice par ce terroriste immigré tunisien, islamiste radical. La France veut aujourd'hui déclarer la guerre à l'islamisme politique, qui entend détruire nos valeurs, nos libertés et notre civilisation. Mais la France se donne-t-elle vraiment les moyens de mener cette guerre ? L'immigration n'est pas la cause première du terrorisme, mais les trois derniers attentats que nous venons de vivre nous confirment qu'elle en est l'une des conditions. Il est temps de mettre un terme au désordre migratoire. Tout à fait ! Chaque année, 300 000 personnes, essentiellement issues des pays musulmans, entrent légalement en France, auxquelles il faut ajouter 150 000 demandeurs d'asile.

aux mineurs étrangers isolés ? Très bien ! Êtes-vous prêt à remettre à plat, totalement, le droit des étrangers, pour que nous nous donnions vraiment les moyens d'expulser ?

voire davantage. Je ne ferai pas l'injure au Sénat, ou au Parlement en général, de dénombrer le nombre de textes législatifs qui sont intervenus en la matière, Notre rôle, madame la sénatrice, est de veiller à l'effectivité et à l'application des lois existantes ; et je puis vous dire

des réseaux sociaux, ce support dont se servent les ennemis de la République pour la frapper. En la matière, vous avez tout à fait raison, il faut revoir la réglementation.

bien avant l'odieux attentat de Conflans-Sainte-Honorine, le Président de la République avait annoncé un projet de loi qui, vous le verrez, sera très ambitieux pour renforcer nos outils de lutte contre cet ennemi.

qui se servent de fausses associations et qui s'introduisent dans des mosquées où des imams radicaux prêchent, non pas la religion, mais la haine. Un par un, nous les traquerons

Les mesures sanitaires sont primordiales, n'y revenons pas, mais la fermeture des petits commerces est difficilement compréhensible. Elle va entraîner un drame économique, car ces petits commerces sont à bout de souffle. Malgré les aides, nombre d'entre eux n'y survivront pas. Leur interdire d'ouvrir, c'est encore creuser la dette et alourdir l'addition du chômage partiel. Cette fermeture est aussi un drame humain. Ce sont eux qui, surtout en zone rurale, tissent le lien social. Lorsque l'on sait que 13 millions de Français ne sont pas connectés, le dispositif de n'apparaît en rien comme un substitut. monsieur le Premier ministre, mais aucune étude n'a encore démontré que librairies, coiffeurs ou auto-écoles étaient des clusters, d'autant moins que les commerçants ont investi pour s'adapter à la situation, pour que la distanciation sociale et les gestes barrières y soient toujours respectés. Aujourd'hui, nous avons un débat absurde sur les produits essentiels et non essentiels. La pâte à tartiner est essentielle, pas les livres ! À côté de cela, les sites internet sont ouverts vingt-quatre pour vendre des produits non essentiels. Cela enrichit les GAFA, déjà milliardaires et non contributeurs fiscaux, laissant mourir ceux qui font la vie des centres-bourgs et des centres-villes. loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, le Sénat a fait adopter à l'unanimité un amendement pour que le préfet puisse autoriser l'ouverture des commerces de vente au détail. Ne peut-on pas être un peu plus créatif et éviter une interdiction uniforme ? Ne peut-on pas autoriser les ouvertures des petits commerces en fonction des situations locales ? Ne peut-on pas autoriser les ouvertures selon des mesures plus fines, avec, par exemple, des prises

Les entreprises de moins de 50 salariés des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie-restauration, de l'événementiel, de la culture, du sport et des secteurs liés, qui ne sont pas fermés administrativement, mais qui enregistrent une baisse de chiffre d'affaires de plus de 50 %, bénéficieront également de cette indemnisation mensuelle, pouvant aller jusqu'à 10 000 euros. Toutes les autres entreprises de moins de 50 salariés subissant une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % bénéficieront d'une aide pouvant aller jusqu'à 1 500 euros par mois. J'ai évoqué le fait que l'activité liée au ne serait pas prise en compte dans l'évaluation du chiffre d'affaires. On peut donc dégager du bénéfice supplémentaire. Je tiens également à mentionner la suppression des cotisations sociales. Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement bénéficieront d'une suppression totale de leurs cotisations sociales. Toutes les PME du tourisme, de l'événementiel, de la culture, du sport et des secteurs liés, qui restent ouverts, mais qui enregistrent une perte de 50 % de leur chiffre d'affaires, auront droit à cette même suppression de leurs cotisations sociales, patronales et salariales. Pour tous les travailleurs indépendants, les prélèvements sont automatiquement suspendus, sans aucune démarche à faire, et les travailleurs indépendants fermés administrativement bénéficieront d'une exonération totale de leurs charges sociales. Je rappelle que le prêt garanti par l'État, le PGE, peut désormais être contracté jusqu'au 30 juin 2021, au lieu du 31 décembre 2020, et que l'État pourra accorder des prêts directs si certaines entreprises ne trouvent aucune solution de financement. Enfin, sur la question des loyers, tout bailleur qui, sur les trois mois d'octobre, novembre et décembre, accepte de renoncer à au moins un mois de loyer, pourra bénéficier d'un crédit d'impôt de 30 % du montant des loyers abandonnés.

et les petits commerces de proximité, comme le montre le cas du géant Amazon. De fait, jamais l'écart entre les petits commerces et ces géants technologiques n'aura été aussi grand.

pour atteindre le chiffre astronomique de 1 650 milliards de dollars, l'équivalent du produit intérieur brut de la Russie- excusez du peu ! La fermeture imposée aux commerces de proximité va encore aggraver une situation de concurrence déloyale. Mais l'autre scandale réside dans les pratiques fiscales d'Amazon, qui ont été décrites comme les plus agressives des entreprises du numérique. Grâce à des montages savants illégaux, accordés par nos amis du Luxembourg, près des trois quarts des bénéfices d'Amazon ne subissent aucune imposition. Cette situation est tout à fait inacceptable, plus encore au moment où les États manquent de moyens financiers pour faire face aux conséquences dramatiques de la pandémie. Il est urgent de mener une bataille au plan international, pour, enfin, taxer de manière effective les GAFA. Au premier trimestre de cette année, les rentes d'Amazon ont augmenté de 26 %. Nous proposons qu'une disposition soit adoptée, dès le budget pour 2021- texte actuellement en discussion au Parlement -, visant à instituer une taxe exceptionnelle sur les bénéfices d'Amazon. Les fonds ainsi récoltés viendraient alimenter un plan d'aide d'urgence aux commerces touchés, notamment aux librairies indépendantes. Je conclurai mon propos avec cette citation de Victor Hugo : « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le faire.

et de la fonction publiques, le 13 octobre dernier, vous annonciez avec le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, un appel à candidatures pour recruter trente « sous-préfets à la relance », afin d'accompagner les citoyens, les élus et les entreprises dans le cadre du plan de relance national pour

Alors que nous entamons l'examen des crédits du projet de loi de finances pour 2021, je tiens à saluer cette initiative, visant à mieux piloter l'ensemble des dispositifs mis en oeuvre par le Gouvernement. Vous décriviez ainsi l'objectif de cette mission prioritaire

Relance comporte trois grands volets : 30 milliards d'euros pour la transition écologique, 34 milliards d'euros pour la compétitivité et la souveraineté économique et 36 milliards d'euros pour la cohésion sociale et territoriale. Ces hauts fonctionnaires s'assureront que ce plan de relance, de 100 milliards sur deux ans, se concrétise bien sur le terrain, c'est-à-dire permette de reconstruire le tissu économique local, l'attractivité de nos territoires et le maillage territorial de l'État. Il s'agit de renforcer l'efficacité de l'État dans les territoires et d'accompagner au mieux les élus et les acteurs territoriaux oeuvrant déjà au quotidien pour mettre en place ces mesures de relance. Loin d'une conception jacobine de l'État, les collectivités territoriales sont placées au coeur de ce plan. En effet, il faut réarmer nos territoires pour que l'État soit un acteur de proximité, qui répond au mieux aux problématiques de nos concitoyens. quels indicateurs ont été mis en place pour choisir les départements dans lesquels seront déployés les sous-préfets à la relance ? Quels sont les critères de réussite de leurs missions ? Où en est-on de leur déploiement ? La parole

Effectivement, il n'y a pas de relance sans simplification, et il ne peut y avoir de simplification si nous ne partons pas du terrain. Nous ne ferons pas la relance depuis Paris, à coups de milliards d'euros ; nous la ferons au plus près des besoins des Français, là où ils vivent. C'est pourquoi le Premier ministre a souhaité que chaque département dispose d'un « chef de projet » dans ce domaine, un sous-préfet à la relance. Pourquoi un sous-préfet ? Vous savez très bien, mesdames, messieurs les sénateurs, les sous-préfets réunissent chaque jour les élus, les chefs d'entreprise et tous les acteurs de terrain. Bref, ils prennent des décisions au bon niveau et nous aident à avancer. À l'heure du second confinement, nous n'avons pas le droit à l'erreur, et l'État, dans tous les territoires, a besoin de renfort.

au plus près du terrain, partout en France, que les milliards d'euros que vous votez deviennent une réalité ! La parole

des interventions ? Quelle est la place de l'équipe médicale dans la décision ? Par ailleurs, pouvez-vous nous donner la capacité actuelle des lits opérationnels, à la fois dans les

ont été fixés, par le ministre, dans un courrier datant du 28 octobre dernier. La méthode a été généralisée à l'ensemble du territoire, avec le déclenchement des premiers paliers de déprogrammation et du plan blanc pour libérer des lits. Dans les régions les plus en tension, toutes les activités chirurgicales, y compris ambulatoires, et médicales pouvant l'être doivent être déprogrammées, dès lors qu'elles mobilisent des ressources humaines pouvant être mobilisées dans les services dédiés

soutenues par des analyses bénéfices-risques de chaque situation. Quand elles sont décidées, elles le sont tout en garantissant que les patients atteints d'un certain nombre de pathologies définies comme « prioritaires » par le ministre- cancers, patients en attente de greffe, patients suivis pour maladies chroniques et requérant des soins urgents, ou encore

Je pense aux extras, aux « permittents », aux bénéficiaires de contrats à durée déterminée d'usage. Je parle des guides-conférenciers, des maîtres d'hôtel, des cuisiniers, des livreurs, des serveurs, des hôtesses, des chauffeurs, des agents d'entretien et de sécurité, et de tous ceux que je ne peux pas citer. Ce sont près de 1 200 000 salariés, typiquement ceux qui étaient menacés par la réforme de l'assurance chômage

a reporté l'entrée en vigueur de ces mesures pour ceux qui sont privés d'emploi depuis le 1 août. Mais la spécificité du travail de certains saisonniers fait qu'ils n'ont pu reprendre leur activité à cause du premier confinement. Ils n'ont donc pas pu recharger leurs droits, du fait de cette réforme, et se trouvent sans solution, si ce n'est celle des minima sociaux. Quant aux autres, ils subiront forcément de plein fouet les effets de ces dispositions : comme ils sont dans l'impossibilité de travailler actuellement, ils n'auront donc aucun droit à recharger. Monsieur le secrétaire nous parlons là de plus d'un million de personnes, qui appellent au secours et que personne n'entend. Je vous pose donc deux questions. Allez-vous consentir à travailler sur une solution de type « année blanche comme pour les intermittents du spectacle, qui permettrait d'attribuer à ces extras et permittents un revenu de substitution ? Allez-vous, enfin, annoncer la suppression de votre réforme de l'assurance chômage ?

Lubin, d'avoir reconnu le travail et l'engagement du Gouvernement pour protéger les plus vulnérables et les plus modestes de notre société face à la crise sanitaire.

d'euros. Sur le fond, vous m'interrogez sur la réforme de l'assurance chômage et sur la façon dont chacun pourra acquérir des droits. Comme vous l'avez indiqué, cette transformation structurelle de notre système d'indemnisation chômage a été repoussée.

le Gouvernement étant particulièrement attentif à la situation de ces Françaises et de ces Français. La parole

monsieur le Premier ministre, vous avez fondé la totalité de la gestion de cette crise sur un seul critère : éviter la saturation des hôpitaux.

avez choisi comme seul paramètre de gestion de cette épidémie l'engorgement des hôpitaux, pourquoi les leçons de la première vague ne vous ont-elles pas servi ? Pourquoi des lits de réanimation n'ont-ils pas été ouverts en nombre suffisant depuis le premier confinement

Depuis le début de la crise, nous avons formé 7 000 professionnels de santé pour qu'ils puissent agir dans les services de réanimation, et je veux ici saluer leur engagement.

Pourquoi aucun lien n'est noué entre les hôpitaux publics et les cliniques privées ? La vérité, monsieur le Premier ministre, c'est que, si vous aviez bien géré l'après-première vague, nous n'aurions pas à connaître un deuxième confinement ! Et je ne peux accepter que, à cause de votre entêtement, nous en connaissions, croyez-moi, un troisième, un quatrième et, peut-être, un cinquième Union Centriste. Monsieur le Premier ministre, notre pays vit des heures graves. En même temps que les attentats et la pandémie, c'est la crise économique et sociale qu'il nous faut combattre. La pauvreté progresse ; un nombre croissant de Français bascule dans la précarité. Après le travail, c'est la perte du logement qui inquiète. Pourrais-je payer mon loyer ? Pourrais-je loger ma famille et mes enfants ? Voilà les questions qui nous sont posées, à nous parlementaires de terrain. Dans ce domaine, aussi, nos compatriotes ont besoin d'être rassurés et protégés. Monsieur le Premier ministre, comme la sécurité sociale, le logement, particulièrement le 1 % Logement, devenu Action Logement, fait partie du pacte social que nous avons hérité de la Résistance et de l'après-guerre. Cet héritage est le fruit d'une triple volonté : garantir et sanctuariser, chaque année, des moyens financiers au logement, y compris dans les périodes difficiles ; gérer ces sommes de manière paritaire, entre patrons et salariés ; mener des actions complémentaires à celles de l'État, dans un esprit de responsabilité sociale pour tous les Français, à commencer par les plus modestes. Ce modèle, ce n'est pas quelque chose du passé qui, sous des prétextes techniques, devrait être abandonné. C'est un modèle pour aujourd'hui, un modèle d'union nationale pour une France qui donne ses chances à chacun. Dans le moment historique que nous vivons, monsieur le Premier ministre, quelles sont les intentions de votre gouvernement en matière de logement, en particulier à l'égard du pilier de notre modèle social

Pour autant, il paraît important de moderniser le fonctionnement et la gouvernance de ce groupe, tout en maintenant sa gestion paritaire. La réforme engagée en 2016 n'a pas été menée à son terme : demeurent d'importants dysfonctionnements d'organisation et d'exécution. Cette réforme permettra également de clarifier la répartition des rôles entre l'État et Action Logement, tout en améliorant la lisibilité et l'efficience des interventions déployées en faveur des citoyens et des entreprises. Vous le savez, le Gouvernement privilégie la concertation avec les partenaires sociaux pour définir des évolutions, les mettre en oeuvre et les contractualiser. Cette Cette concertation a d'ores et déjà commencé. D'ailleurs, l'ensemble des partenaires sociaux seront reçus, dès demain, par Élisabeth Borne, Emmanuelle Wargon et Olivier Dussopt. Ces discussions ont vocation à aboutir au printemps de 2021.

au moment où- on le sait bien -ce sujet va être majeur La parole est à M. Vincent Segouin, pour le groupe Les Républicains. Les Républicains. Monsieur le ministre, la question que je vais poser n'est pas la mienne, mais celle de centaines de personnes- élus locaux, commerçants ou indépendants -à qui j'ai eu l'occasion de parler au téléphone ces derniers jours. je dis bien tous, sont dans une situation désespérée : ils n'attendent rien de bon pour leur activité, et leur existence vire parfois au drame. Plusieurs maires m'ont ainsi parlé de cas de détresse psychologique chez les commerçants de leur commune.

! Plus je vous écoute, plus votre manque de cohérence me désespère. On laisse les grandes surfaces ouvertes, mais, en même temps, on ferme les petits commerces, qui pourtant respectent les mesures sanitaires. On ferme nos restaurants, mais, en même temps, on laisse ouverts des restaurants d'entreprise et des cantines à grande fréquentation. On empêche les gens d'aller chez le libraire, mais, en même temps, on les laisse se masser dans les transports en commun. On interdit les coiffeurs à domicile, mais, en même temps, on autorise les livraisons ou les travaux à domicile. On laisse les gens passer les frontières de notre pays sans aucun contrôle, mais, en même temps,

le président Erdogan multiplie les menaces contre la France, comme il l'avait d'ailleurs fait ces derniers mois contre le gouvernement autrichien. Tout à fait ! Sa politique impérialiste se manifeste en Méditerranée, en Libye, en Syrie, en Irak et, désormais, dans le Caucase, où il soutient concrètement l'offensive de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Nous soutenons la position claire et ferme du Président de la République, non pas contre le peuple turc, à qui nous exprimons notre solidarité après le tremblement de terre d'Izmir, mais contre un pouvoir autoritaire, qui menace la stabilité de la région et la sécurité de l'Europe, ... Tout à fait ! ... alors même qu'il est membre de Monsieur le ministre, il faut maintenant que les actes soient à la hauteur des paroles. La France va-t-elle vraiment demander des sanctions financières contre la Turquie ? Alors que son processus d'adhésion à l'Union européenne est au point mort, ce pays perçoit-il encore des fonds de préadhésion ? Le boycott des produits français est décrété en violation de l'union douanière entre l'Europe et la Turquie. S'il perdurait, seriez-vous prêt à demander sa suspension ? En septembre dernier, un rapport de l'ONU a dévoilé les exactions très graves commises à l'encontre des Kurdes de Syrie : quelles suites envisagez-vous d'y donner ? Comptez-vous saisir le Conseil de sécurité des Nations unies ? Pouvez-vous d'ailleurs nous garantir que la France a mis un terme à toute vente de matériel militaire à la Turquie ? Enfin, après la nécessaire dissolution de l'organisation extrémiste des Loups gris, comptez-vous agir résolument contre l'influence du régime turc sur le territoire national ?

majeurs. Mais, ces dernières semaines, nous avons franchi dans nos relations avec la Turquie un palier inadmissible entre pays alliés. Les insultes, les calomnies, la volonté d'instiller une campagne de haine contre la France et l'Europe sont de nature totalement différente : ce sont des menaces. Nous attendons que le président turc et son gouvernement y mettent un terme immédiat. Nous ne tolérerons

qu'elle soit nationale ou européenne. Contrairement à d'autres secteurs largement délocalisés, les industries de défense françaises continuent à produire en France et pèsent dans notre économie. Engagées au service de la sécurité collective, elles représentent un vivier de compétences rares et d'emplois dans les territoires. Cette excellence permet à nos armées de disposer de la meilleure technologie possible pour conserver la supériorité sur le terrain. Elle bénéficie également au commerce extérieur, en permettant de rivaliser à l'export avec les pays à bas coûts. Pour autant, le secteur de la défense n'est pas exempt de fragilités et les confinements de l'année 2020 vont laisser des traces. Vous le savez, les entreprises françaises de technologies sensibles suscitent déjà les convoitises. elles sont passées sous contrôle étranger. J'ai également évoqué le cas de Photonis, l'un des leaders mondiaux de la vision nocturne, qui, après maintes péripéties et interventions de l'État, serait sur le point d'être racheté par un groupe américain.

pays est face à un risque de pénurie de sang, dû tout autant aux difficultés actuelles de collecte qu'à la non-revalorisation des personnels de l'Établissement français du sang, sang, l'EFS. Nous avons besoin de 10 000 dons par jour pour satisfaire aux soins de 1 million de malades chaque année. Or la crise sanitaire entrave considérablement la collecte moins de dons de la part des étudiants, qui figurent parmi les populations les plus généreuses en la matière, et moins de personnel dans les entreprises, où ont lieu nombre de collectes. En parallèle, les professionnels de l'EFS sont eux aussi touchés par le virus et nombre de bénévoles sont empêchés pour cause de vulnérabilité.

ressentent un profond sentiment d'injustice. Eux aussi sont au front, depuis longtemps, et plus encore depuis la crise sanitaire. Monsieur le ministre, allez-vous revaloriser le statut des personnels de l'EFS ? Comment comptez-vous agir et réagir

et, dès lors, reposent sur le don régulier de sang, de plaquettes ou de plasma. Je pense notamment à la prise en charge des effets de certaines pathologies de longue durée, comme les cancers ou les maladies du sang.

La séance est reprise. Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande que l'examen en nouvelle lecture du projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire se poursuive le jeudi 5 novembre au soir. Acte est donné de cette demande. Nous pourrions fixer le début de la discussion générale sur ce texte demain à dix-neuf heures. La commission se réunirait pour examiner les amendements de séance durant la suspension de séance, et nous entamerions l'examen des articles à la reprise du soir. Enfin, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance serait fixé à l'ouverture de la discussion générale. Y a-t-il des observations ? ... Il en est ainsi décidé. Par ailleurs, par courrier en date du mardi 3 novembre, M. Claude Malhuret, président du groupe Les Indépendants - République et territoires, demande l'inscription à l'ordre du jour de l'espace réservé à son groupe du jeudi 19 novembre de deux débats intitulés La forêt française face aux défis climatiques, économiques et sociétaux » et « Contenus haineux sur internet : en ligne ou hors ligne, la loi doit être la même ». Acte est donné de cette demande. J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030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

et échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'État du Qatar et de l'accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l'adoption de ce texte. L'ordre du

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde relatif à la prévention de la consommation illicite et à la réduction du trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chimiques, et des délits connexes

Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les crises sanitaire et sécuritaire que nous traversons ont démontré l'importance de répondre avec la plus grande détermination au problème mondial de la drogue.

cette pandémie a accru la vulnérabilité des usagers, qui ont connu des difficultés pour accéder au dispositif de soins ou, parfois, se sont tournés vers des substances ou des modes de consommation plus nocifs. La fin de la crise sanitaire, quel que soit son horizon, ne résoudra pas ces difficultés, bien au contraire, avec la circulation des stocks de drogue surnuméraires n'ayant pu être écoulés et l'existence de publics encore plus fragilisés. Alors que les trafics de stupéfiants ne cessent de s'étendre à l'échelle mondiale, notre réponse doit, aujourd'hui plus encore, passer par une action coordonnée à l'échelle internationale. fait, ces trafics constituent un phénomène véritablement mondial, qui se joue entre pays de production, de transit et de destination. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres pour agir à la fois en amont, afin d'éviter que nos populations, en particulier les personnes les plus vulnérables, ne tombent dans l'addiction, et en aval, pour offrir une voie de sortie de la dépendance à ceux qui le souhaitent, suivant une approche respectueuse des droits humains.

depuis 1998 par un partenariat stratégique, dans le cadre duquel se sont développées des coopérations ambitieuses dans les domaines de la défense, de l'espace, de la sécurité ou encore du climat. L'accord intergouvernemental relatif à la prévention de la consommation illicite et à la réduction du trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chimiques, et des délits connexes,

ensuite, en tant qu'acteur constructif de la scène internationale en matière de lutte contre les produits stupéfiants et en tant que soutien de notre approche équilibrée faisant droit aussi bien aux impératifs de la lutte contre les trafics qu'à la nécessité de mener des politiques de prévention. L'Inde doit être associée à cette lutte. Face à la double pression exercée par les pays les plus laxistes, désireux notamment de légaliser largement l'usage des drogues, et les plus fermés, promoteurs d'une réponse exclusivement répressive, donc incomplète, l'Inde est un soutien essentiel pour la préservation de ce cadre international.

que peut faire peser sur notre sécurité nationale la situation spécifique de ce pays de plus de 1,3 milliard d'habitants, qui est à la fois une zone de transit, de production et de consommation de stupéfiants. Située à l'interface de plusieurs zones majeures de production, l'Inde est un pays de transit de ces produits vers le monde entier, qu'il s'agisse de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique du Nord ou même de l'Asie du Sud-Est. Ce renforcement de notre coopération est d'autant plus nécessaire que la question des drogues, je le rappelle, a partie liée avec le terrorisme. De fait, le trafic de stupéfiants constitue, toujours plus, l'une des premières sources de revenus des réseaux terroristes islamistes mondiaux opérant notamment dans le sous-continent indien, en particulier en Afghanistan. Afghanistan. Par ailleurs, l'Inde est devenue un lieu de production de différents stupéfiants et précurseurs chimiques, exportés vers des marchés étrangers où leur consommation provoque, vous le savez, des difficultés sanitaires majeures au sein des populations de nos pays. Enfin, la croissance de la consommation de drogues en Inde doit nous alerter, compte tenu de ses conséquences sur la santé publique dans ce pays, comme sur le développement accru de réseaux criminels. à votre approbation, le premier engagement juridiquement contraignant conclu avec l'Inde en matière de coopération policière et judiciaire, constitue un jalon essentiel pour nous permettre d'atteindre l'ensemble de ces objectifs.

les champs de coopération renforcée qu'il ouvre permettront à la fois une montée en puissance de notre action commune en matière de lutte contre la consommation et le trafic de stupéfiants et une meilleure prise en compte dans nos échanges de l'ensemble des enjeux sanitaires et sociaux. Ainsi, cet accord permettra d'encourager le développement d'actions de coopération visant à réduire effectivement la production de stupéfiants, notamment de précurseurs chimiques, ainsi que leur éventuel trafic entre nos deux pays et au-delà. Il nous donnera également les moyens d'agir sur la demande, en promouvant auprès de nos partenaires indiens notre approche en matière de prévention de la consommation de drogues. Là aussi, cela passera par la conduite nouvelle d'actions conjointes d'éducation et de sensibilisation des publics les plus vulnérables.

en fixant un socle d'obligations et de garanties fondamentales précises en matière de protection des données personnelles, en deçà duquel aucune opération de traitement ou de transfert de données ne pourra être effectuée.

voulue par le Président de la République, de renforcement de notre relation bilatérale avec l'Inde, notamment sur les questions stratégiques et de sécurité.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la France entretient avec l'Inde une relation bilatérale ancienne, fondée sur la confiance et le partage de valeurs communes. Cette relation s'est enrichie ces dernières années, avec la multiplication de rencontres de haut niveau. l'Inde et la France ont conclu un partenariat stratégique global, qui a mis en place une coopération étroite dans les secteurs de la diplomatie de la défense. Il s'est traduit par la conclusion, en 2016, d'un contrat d'acquisition de trente-six avions de combat Rafale, dont le premier a été livré en octobre 2019. Notre coopération est intense dans les domaines de la sécurité, du nucléaire civil et de l'énergie. Un dialogue stratégique réunit les deux parties au plus haut niveau deux fois par an. L'Inde occupe une place importante dans la stratégie de défense française en Indopacifique. S'agissant de la lutte contre les trafics de drogue, l'Inde y prend une part active, en participant aux travaux de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, ainsi qu'à l'initiative du Pacte de Paris, lancée en 2003 pour lutter contre le trafic d'opiacés en provenance d'Afghanistan. Compte tenu de son poids démographique et de son positionnement géographique, l'Inde est un acteur régional majeur de la lutte contre les flux illicites de produits stupéfiants, dont elle est à la fois un pays de consommation, de transit et de production. Comme en France, on y observe une augmentation de la consommation de drogues, qu'il s'agisse d'héroïne, d'opioïdes détournés de leur usage médical ou encore de cannabis. De par sa situation à proximité du Triangle d'or et surtout du Croissant d'or, zone de production d'opium la plus importante au monde, l'Inde est l'une des principales routes pour le trafic international d'héroïne à destination de la Chine et de l'Asie du Sud-Est, mais aussi de l'Australie et de l'Amérique du Nord. L'Inde se situe aussi sur la route sud par laquelle transiteraient environ 10 % des opiacés à destination de l'Europe et de la France. Enfin, l'Inde, deuxième leader mondial des médicaments génériques derrière la Chine, avec 20 milliards de dollars d'exportations annuelles cette année, connaît de nombreux détournements de médicaments par des organisations criminelles. Sont concernés notamment l'éphédrine et certains antalgiques, comme le Tramadol, qui sont consommés comme drogues, sans parler des médicaments contrefaits par des entreprises installées sur le territoire indien. Cet accord bilatéral est le premier engagement juridiquement contraignant conclu avec l'Inde en matière de coopération policière. Il s'agit d'un accord sectoriel, portant exclusivement sur la prévention de la consommation illicite et la réduction du trafic illicite de stupéfiants. sera mis en oeuvre en parfaite cohérence avec les engagements bilatéraux liant nos deux États dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale et d'extradition : la convention bilatérale d'entraide judiciaire pénale du 25 janvier 1988 et la convention bilatérale d'extradition du 24 janvier 2003. La commission s'est naturellement penchée avec la plus grande attention sur l'applicabilité de la peine de mort, proscrite par notre Constitution, La convention d'extradition de 2003 permet déjà expressément à la France de refuser la remise d'un individu demandée par l'Inde en l'absence de garantie que la peine de mort ne sera pas prononcée, exécutée. Comme l'accord d'entraide judiciaire de 1988, l'accord que nous examinons aujourd'hui contient des dispositions supplémentaires permettant, comme M. le secrétaire d'État l'a expliqué, d'opposer un refus aux demandes de coopération si elles devaient aboutir à l'exécution de la peine capitale en l'absence même de toute clause expresse, l'ordre public français et les engagements internationaux de la France s'opposent à ce que notre pays puisse apporter son aide en matière pénale aux États dans lesquels une personne mise en cause est exposée à la peine capitale ou à des traitements inhumains ou dégradants. Quant aux stipulations relatives à la protection des données personnelles, elles apportent un haut niveau de garantie, dans la mesure où la communication de ces données aura lieu dans le strict respect de la législation nationale et des procédures définies par le droit interne. En outre, les échanges d'informations prévus par le présent accord ne seront pas, par nature, liés à une enquête spécifique en cours ou à un dossier relatif à une personne en particulier, mais porteront davantage, s'agissant de la coopération opérationnelle, sur la structure d'une organisation criminelle, son mode opératoire ou les techniques de blanchiment d'argent. Cet accord de coopération nous a semblé un instrument utile dans la lutte contre le trafic de drogue. Son approbation est attendue par les services des ministères des affaires étrangères, de l'intérieur et de la justice. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous invite à adopter le projet de loi qui nous est soumis. La parole

Si les produits stupéfiants sont dangereux pour la santé de ceux qui les consomment, leurs trafics sont néfastes, plus généralement, pour l'ensemble de la société. En effet, ces produits font l'objet d'un commerce lucratif dont les fonds viennent alimenter d'autres activités criminelles, au premier rang desquelles le terrorisme. les liens entre la culture afghane du pavot et le financement des talibans ne sont plus à démontrer- non plus que ceux qui unissent les productions du Triangle d'or aux mafias et guérillas de cette région. Parce que le trafic de drogue ne connaît pas de frontières, parce qu'il participe au financement d'actions de déstabilisation contre les États, ces derniers ont intérêt à unir leurs moyens dans leur combat contre la drogue, comme M. le secrétaire en raison notamment de sa situation géographique, qui la place au carrefour de nombreux trafics, est d'ores et déjà un des acteurs incontournables de la lutte antidrogue. à notre approbation cet après-midi vise à améliorer la coopération policière entre nos deux pays dans ce domaine. Je fais partie des voix qui se sont élevées pour alerter sur le risque potentiel que comporterait cet accord. De fait, l'Inde applique la peine de mort à l'encontre des auteurs de certaines infractions relatives aux stupéfiants. relatives aux stupéfiants. La France n'enfreindrait-elle pas ses engagements abolitionnistes en coopérant avec un pays qui, sur la base de cette coopération, pourrait condamner des individus

mettant en danger la vie de nos concitoyens. Chaque État est souverain : il décide donc souverainement des règles qu'il souhaite établir. Il n'appartient à personne de dire à l'Inde, État souverain et démocratie de plus de 1,353 milliard de personnes, ce qu'elle devrait ou ne devrait pas faire. L'Inde et la France luttent toutes deux contre le trafic de drogue et peuvent envisager de coopérer dans ce domaine, dans le respect de la souveraineté de nos deux pays. nous devons analyser cet accord en nous assurant qu'il ne contribue pas à faire concourir la France, par ce canal, à l'exécution de peines capitales. En effet, les engagements de notre pays l'obligent à abandonner une coopération lorsque la peine de mort est envisagée à l'encontre de personnes mises en cause. Ce principe est inscrit dans les accords relatifs à la coopération judiciaire et l'extradition.

En pratique, cet accord favorisera l'échange d'informations entre la France et l'Inde. Compte tenu de la croissance des trafics illicites de stupéfiants et de la position stratégique de l'Inde, l'objectif peut se comprendre, même si des accords multilatéraux existent en la matière. Si le groupe écologiste a demandé le retour à la procédure normale pour l'examen de ce projet de loi, c'est parce que ce dispositif nous inquiète : de fait, nous trouvons pour le moins curieux qu'il ne fasse pas plus débat ... L'absence de toute mention relative à la peine de mort dans un projet d'accord avec un pays qui applique encore la peine capitale en matière de trafic de stupéfiants est incompréhensible

il n'énonce nullement qu'une mention ne serait exigée que pour les accords relatifs à la remise des personnes. Cette décision exclut l'extradition d'une personne vers un pays où la peine de mort est prononcée, dès lors qu'aucune convention ne vient l'exclure ; aucune autre question de droit ne lui était posée. droit ne lui était posée. En l'occurrence, ne pas prévoir que la remise de renseignements puisse permettre de condamner une personne à la peine de mort entraîne la violation par la France de ses obligations positives à l'égard de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, il n'est pas compréhensible que, politiquement, il ne soit pas possible d'exiger une telle garantie de l'Inde, alors que la France l'a exigée des États-Unis pour ratifier le traité d'extradition du 23 avril 1996. Les organisations de défense des droits humains, au premier rang desquelles la Ligue des droits de l'homme, ont réussi à alerter le Sénat. À la suite de cette interpellation, monsieur le rapporteur, vous évoquez deux garde-fous,

Il est à ce titre curieux, monsieur le secrétaire d'État, que dans l'étude d'impact, ni la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne soient mentionnés parmi les engagements internationaux que la France doit respecter.

avant éventuellement de refuser de donner un renseignement. Le dossier entier n'est bien sûr pas envoyé et se poserait alors un problème de traduction. Il est évident que cela ne se fera jamais. L'examen au cas par cas, pour envisager si la peine de mort pourrait être prononcée pour chaque renseignement demandé, et le blocage en conséquence de la transmission d'informations sont totalement illusoires.

Compte tenu des inquiétudes que suscite ce texte, monsieur le secrétaire d'État, je conclus mon propos en vous demandant de renégocier cet accord. La République de l'Inde doit s'engager à ne pas prononcer de condamnation à mort dès lors que la France a contribué de quelque manière que ce soit à la résolution d'une affaire. Cela doit figurer noir sur blanc.

sérieuses ! De plus, l'industrie pharmaceutique indienne, qui est championne du monde en matière de contrefaçon, fabrique toute une série de produits pharmaceutiques qui sont exportés vers l'Europe et vers les États-Unis,

La lutte contre ce fléau nécessite une coopération très étroite reposant sur l'échange d'expertises, l'échange d'informations et la formation d'agents spécialisés.

L'étude d'impact annexée au projet de loi évoque le lien entre un médicament fréquemment détourné de son usage, le Tramadol, et le financement des groupes terroristes en Afrique et dans d'autres pays du monde. accord est susceptible d'ouvrir la voie à un renforcement de la lutte contre la contrefaçon de médicaments.

la loi indienne relative aux stupéfiants et aux psychotropes prévoit la possibilité de condamner à mort une personne pour trafic de stupéfiants. Il faut toutefois espérer

peine de mort, la France doit continuer à appeler l'Inde à observer ce moratoire en vue de l'abolition définitive de la peine de mort.

L'accord que nous devons approuver aujourd'hui porte sur la prévention et la réduction du trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chimiques. Le sujet est grave et mérite notre attention. Les chiffres sont inquiétants la consommation mondiale de drogue augmente. Cette augmentation n'épargne ni la France ni l'Inde. L'essor de la toxicomanie est notamment lié à l'accroissement des réseaux criminels qui s'adonnent au trafic de stupéfiants. Derrière chaque trafic local, derrière chaque consommateur isolé se trouve au départ un réseau international. Combattre le fléau de la drogue implique donc de s'attaquer à chacun de ses maillages. de ses maillages. Si l'Inde n'est pas l'un des pays les plus stratégiques dans la lutte contre le trafic de stupéfiants- elle n'est pas identifiée comme la source immédiate et directe de trafics en France -, il n'en demeure pas moins que, par sa taille et son important bassin de population, elle est fortement touchée par la consommation de stupéfiants. Plus encore, par son positionnement géographique, elle est un point de passage, dans la région, entre les réseaux du croissant du croissant d'or- Afghanistan, Iran et Pakistan -et du triangle d'or au confluent du Laos, de la Birmanie et de la Thaïlande. De ce point de vue, l'Inde joue un rôle actif dans la lutte internationale contre les drogues, l'efficacité de son action étant l'une des conditions d'une meilleure répression du trafic. doit viser aussi bien les stupéfiants les plus traditionnels que le détournement des médicaments ou des molécules servant de matière première à la production de drogues. Un tel combat sera d'autant plus bénéfique que le

le Gouvernement présentait à Marseille le 17 septembre 2019 un Plan national de lutte contre les stupéfiants, qui fixait une liste de six objectifs, dont le développement de la coopération internationale. L'accord discuté aujourd'hui y participe pleinement, en élargissant les modalités de coopération technique et opérationnelle entre l'Inde et la France. Dans un premier temps, s'agissant de la coopération technique, cet accord contribuera indéniablement à permettre une meilleure compréhension des réseaux de trafiquants,

Il faut faciliter les échanges juridiques, les formations et les échanges d'expertise. Toutefois, l'information ne suffit pas. Dans un second temps, il faut agir et se donner les moyens de l'action.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'accord entre la France et l'Inde qui nous est soumis doit être examiné d'un double point de vue la pertinence de mesures de coopération renforcée pour lutter contre le trafic de stupéfiants, d'autre part, celui des conditions concrètes de cette coopération avec le régime politique actuel de ce pays, un régime extrémiste hindouiste raciste, foulant aux pieds les droits fondamentaux, notamment ceux des citoyens indiens musulmans et chrétiens. Au nom

C'est l'une des raisons de notre inquiétude sur les possibles conséquences en matière de droits humains de l'application de cette convention. L'objet de ce texte est de se donner de nouveaux moyens de lutte contre le trafic de produits stupéfiants, fléau indéniable et de grande ampleur. l'Inde est bien l'une des plaques tournantes du trafic mondial d'opiacés. Elle est par ailleurs le premier producteur mondial de médicaments génériques- la France est d'ailleurs une très bonne cliente de l'Inde, notre pays ne produisant que 5 % de la consommation médicinale nationale.

L'Inde est aussi le théâtre d'un véritable trafic d'éphédrine et de Tramadol. Enfin, il faut souligner les liens structurels- ils sont de plus en plus documentés -entre tous les types de trafics transnationaux, par exemple ceux de produits stupéfiants, les réseaux de blanchiment

que les Européens dépensaient au moins 24 milliards d'euros par an en drogues et produits stupéfiants. La convention pourrait donc renforcer un indispensable effort de coordination et de coopération dans la lutte contre ces trafics, dans l'esprit des travaux de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime et du pacte de Paris de 2003. La coopération avec l'Inde appelle toutefois de lourdes remarques, au moment où le régime de Modi foule aux pieds l'État de droit au nom de théories ouvertement racistes, où les milices armées d'extrême droite hindouiste perpètrent des massacres dans ce pays et où la destination financière des trafics visés par la convention doit être interrogée, y compris dans les rangs du régime de New Delhi. Pouvons-nous fermer les yeux sur l'état du système sur l'état du système judiciaire et policier de ce pays et sur le possible recours par ce régime à la peine de mort, contraire aux conventions internationales dont la France est signataire Notre vote contre en commission tendait à alerter sur ces enjeux essentiels. Nous avons entendu les réponses du Gouvernement : la convention devant servir à échanger des informations structurelles sur les réseaux, et non sur les personnes, les risques d'une condamnation à mort d'une personne poursuivie du fait de la transmission d'informations françaises seraient limités. Quand bien même cela arriverait, ces informations tomberaient sous le coup de la convention d'extradition de 2005, qui contient une clause obligeant l'Inde à renoncer à une exécution. Si l'accord ne contient pas une clause de non-application de la peine de mort, ce qui est à nos yeux profondément regrettable, il instaure, nous dit-on, des garde-fous aux articles 2 et 5 permettant à la France de se soustraire à la coopération lorsqu'elle pressent une entorse possible à ses engagements internationaux.

substances psychotropes et de précurseurs chimiques, et des délits connexes. Cet accord s'inscrit dans une relation bilatérale avec l'Inde, relation qui s'est enrichie ces dernières années par la multiplication de rencontres de haut niveau. De partenaire naturel théorique, l'Inde est devenue l'un des axes déterminants de la stratégie française en Indopacifique.

La chaleur du communiqué de condoléances et de soutien que nous a adressé l'ambassade d'Inde à la suite de l'attentat horrible contre le professeur Samuel Paty et des attaques personnelles inacceptables contre le Président de la République a tranché avec le silence pesant de l'ambassade de Chine. Compte Compte tenu de son poids démographique de 1,3 milliard d'habitants et de son positionnement géographique, l'Inde est un acteur régional majeur de la lutte contre les flux illicites de produits stupéfiants et de faux médicaments. Sa situation la place à proximité du triangle d'or- Laos, Birmanie, Thaïlande -et surtout du croissant d'or- Iran, Afghanistan, Pakistan -, zone de production d'opium la plus importante au monde. L'Inde est l'une des principales routes pour le trafic international d'héroïne, d'héroïne, la route dite Sud par laquelle transiteraient environ 10 % des opiacés à destination de l'Europe et de la France. Les flux illicites de stupéfiants produits en Inde vers la France consistent essentiellement en drogues de synthèse.

c'est le cas de l'éphédrine et de certains antalgiques, comme le Tramadol, qui sont consommés comme drogues, sans parler des médicaments contrefaits par des entreprises installées sur le territoire indien. Comme l'a rappelé notre collègue Hugues Saury en commission lors de l'examen du rapport de ce texte, ce phénomène se traduit par des centaines de milliers de morts chaque année, principalement en Afrique. Ces victimes sont le plus souvent des enfants. Non seulement les médicaments de qualité inférieure ou falsifiés ont un impact tragique pour les malades et leurs familles, mais ils représentent aussi une menace en termes de résistance aux antimicrobiens. Cet accord est nécessaire, parce qu'il constitue une occasion de promouvoir les actions de prévention et de traitement auprès de notre partenaire indien et parce qu'il permettra de combattre de véritables fléaux, notamment sur notre territoire national- le trafic de drogue, les problèmes de santé publique ou même le terrorisme.

fervent abolitionniste de la peine de mort, je souhaite rappeler que, à la différence de son voisin chinois qui exécute environ un millier de personnes chaque année, la Cour suprême de l'Inde a estimé que la peine capitale ne saurait plus être prononcée qu'à titre exceptionnel.

il nous apparaît qu'elles ne sauraient être un argument pour ne pas voter ce texte susceptible de contribuer à sauver de nombreuses vies.

Merci

C'est parce que l'Inde est une grande puissance internationale qui s'inscrit dans le multilatéralisme que la France souhaite renforcer depuis plusieurs années un partenariat stratégique. De leur côté, les autorités indiennes sont de plus en plus favorables à un partenariat solide et durable

C'est à l'aune de cette stratégie et de ce partenariat que nous devons étudier le texte qui nous est présenté aujourd'hui. Celui-ci prévoit le renforcement de la coopération entre la France et l'Inde en matière de lutte contre les stupéfiants et leur consommation illicite dans le cadre de la réduction de ces trafics. de loi prévoit à la fois la conduite d'actions de prévention et de lutte contre le trafic de drogue et de précurseurs chimiques, le contrôle et la surveillance de la production de ces précurseurs, la prévention de la consommation de drogue grâce à des campagnes de sensibilisation et la mise en place de politiques publiques, sanitaires et sociales auprès des personnes concernées.

domaines. Cet accord de prévention de la consommation illicite en vue de la réduction du trafic illicite de stupéfiants s'inscrit en cohérence avec l'initiative du pacte de Paris de 2003, lancée par la France et la Russie pour lutter contre le trafic d'opiacés en provenance d'Afghanistan à l'époque du conflit. Nous savons tous que les produits stupéfiants sont l'une des principales sources de financement des groupes terroristes armés islamistes.

Elle doit aussi combattre le séparatisme au nord-est et gérer la rébellion de l'armée naxalite au centre. Par ailleurs, nous ne pouvons ignorer la progression de la radicalisation à l'échelle régionale. Les attentats de 2016 au Bangladesh et de 2019 au Sri Lanka ainsi que la situation aux Maldives en sont la tragique démonstration. Il est donc primordial d'évaluer à leur juste mesure les articulations entre trafic de drogue, criminalité internationale et terrorisme. Cette porosité entre criminalité et terrorisme doit véritablement être prise en compte. Je rappelle d'ailleurs que la France et l'Inde ont signé en 2003 la convention de Palerme contre la criminalité transnationale. L'accord que nous examinons répond également à une stratégie internationale de lutte contre la drogue et les criminalités qui y sont liées. Il dépasse donc le seul prisme bilatéral franco-indien. L'Inde est une plateforme de transit pour le trafic de drogue de la région et une voisine directe du triangle d'or- Laos, Birmanie, Thaïlande du croissant d'or- Iran, Afghanistan, Pakistan -, qui est la zone de production d'opium la plus importante au monde. Le sous-continent indien est donc l'une des principales routes pour le trafic international d'héroïne vers la Chine, l'Asie du Sud-Est, l'Australie et l'Amérique du Nord, route qui se termine en Europe et en France. En Inde, l'usage récréatif du cannabis est interdit depuis 1985, mais certaines régions, comme le Madhya Pradesh, produisent des volumes atteignant 240 tonnes par an. L'autre problème tient au taux de tétrahydrocannabinol, ou THC, très élevé de ce type de chanvre : les effets sur les consommateurs sont très graves. De plus, dans le contexte actuel où le risque pandémique est quotidien, notre collaboration avec l'Inde dans la lutte contre les produits illicites est primordiale, car ce pays est le second producteur mondial de médicaments génériques. Lutter contre le trafic de produits illicites qui servent de base aux médicaments est un défi pour la santé publique mondiale. En effet, ces produits font l'objet non seulement de trafics, mais aussi de contrefaçons dont les ressorts sont tentaculaires. Selon l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments (Iracm), le trafic de médicaments et de produits les composants est vingt fois plus lucratif que le trafic d'héroïne. En 2013, en Chine, le trafic de médicaments représentait près de 73 milliards de dollars. Pour 10 000 dollars investis, la contrefaçon de médicaments rapporte entre 200 000 dollars et 450 000 dollars. Ces sommes sont à terme blanchies et réinjectées dans l'économie légale. Ainsi, les trafiquants réussissent à pénétrer des circuits légaux le reconditionnement de médicaments. Alors que les États sont très en retard en termes de législation et que les trafiquants font preuve d'une adaptabilité hors norme, cet accord va dans le bon sens. Il représente une avancée significative pour essayer d'endiguer ces pratiques dont les conséquences sont dramatiques en 2013, plus de 122 000 enfants africains sont décédés du fait des contrefaçons médicamenteuses. Mes chers collègues, je tiens aussi à appeler votre attention sur les conséquences des trafics de produits servant à l'élaboration de drogues de synthèse. Ces nouveaux produits de synthèse (NPS) font des ravages chez les jeunes Français et, plus largement, chez les jeunes du monde entier. Des vies sont brisées à la suite de la prise de MDMA, de méthamphétamines, de kétamine un coût humain autant que financier pour le système français. Par ailleurs, les concentrations de ces drogues sont d'autant plus problématiques que leur potentiel addictif est exponentiel.

de la loi de 1985 relative aux stupéfiants et substances psychotropes. Cet article prévoit la possibilité de condamner à mort un individu pour trafic de stupéfiants dans certains cas particulièrement graves impliquant une récidive.

Aussi, j'espère que ce débat et vos réponses, monsieur le secrétaire d'État, permettront d'apporter des explications bienvenues. Pour ma part, je rappelle qu'il a fallu cinq ans pour parvenir à une rédaction qui satisfasse les deux parties. C'est la preuve que la France a été exigeante et qu'elle n'a pas bradé ses idéaux et valeurs. En outre, la convention bilatérale franco-indienne en matière d'extradition du 24 janvier 2003 est explicite sur le risque d'application de la peine de mort

: « Si le fait en raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de l'État requérant et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de l'État requis ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition peut n'être accordée qu'à la condition que l'État requérant donne des assurances jugées suffisantes par l'État requis que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée. » Je veux croire que cet accord représente un bon véhicule pour continuer les échanges constructifs entre nos deux pays et diffuser les valeurs que nous défendons.

en Inde. Je ne redonnerai pas lecture des articles 2 paragraphe 3 et 5 paragraphe 3, qui ont été cités à plusieurs reprises : ils sont extrêmement clairs sur le plein respect de l'intégralité de nos engagements internationaux, en particulier du protocole n° 6 de la Convention européenne

de mon intervention en discussion générale, mais le sujet mérite que l'on s'y attarde. Sur l'initiative de Jacques Chirac, la France a inscrit son opposition à la peine capitale dans la loi fondamentale. Depuis plusieurs décennies, notre pays s'engage pour l'abolition de la peine de mort partout dans le monde. À ce sujet, je me permets de rappeler à notre assemblée que la France a adhéré au deuxième protocole facultatif se rapportant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Ce protocole prévoit notamment la compétence du Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies pour examiner la situation de chaque État concernant le respect de ses obligations. La question de la non-inclusion d'un engagement de l'Inde à ne pas respecter l'interdiction de la peine de mort dans le présent accord signé par la France sera examinée par ce comité. Il y va du rayonnement ce comité. Il y va du rayonnement et de la crédibilité internationale de notre pays. S'agissant de l'Inde, le problème est encore plus grave. En droit indien, la présomption d'innocence en matière de détention de stupéfiants est écartée au profit d'une présomption de culpabilité. C'est au suspect de démontrer qu'il n'a pas commis l'infraction dont on l'accuse. Or la présomption d'innocence fait partie des principes directeurs de la procédure pénale à valeur constitutionnelle, aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et conventionnelle, avec l'article 6 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Est également inclus le droit à un procès équitable. Rappelons-le, il n'est pas loisible aux États contractants de conclure avec d'autres États des accords dont les dispositions sont en conflit avec leurs obligations

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières

Cet accord est clairement imputable au travail de compromis rapidement engagé avec le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Grégory Besson-Moreau, et ses équipes et, bien entendu, à la volonté du ministre de faire aboutir ce texte, « quoiqu'il en coûte » en matière médiatique, si vous me permettez l'expression. Cet état d'esprit qui a permis la coconstruction d'un texte était nécessaire, car la situation était urgente. Il en résulte un texte très clair. D'une part, les néonicotinoïdes demeurent interdits en France ; leur interdiction a d'ailleurs été consolidée juridiquement par le projet de loi. Seule la filière betterave sucrière pourra bénéficier, par arrêté des ministres de la transition écologique et de l'agriculture, de dérogations pour l'usage de semences jusqu'au 1 juillet 2023, soit pour trois campagnes. part, des garanties essentielles pour l'équilibre du projet de loi ont été annoncées lors de la navette parlementaire. Je pense au plan national de recherche et d'innovation pour accélérer la recherche d'alternatives aux néonicotinoïdes, au plan de prévention proposé par la filière et au conseil de surveillance.

légèrement la composition du conseil de surveillance pour le rendre plus efficace. Ne seront ainsi mentionnés dans la loi que les acteurs concernés par la problématique de la culture, et le ministre de la santé y sera associé. Le Gouvernement pourra, s'il le souhaite, ajouter d'autres acteurs.

membres de l'opposition. Ensuite, la procédure de rédaction de l'arrêté de dérogation a été simplifiée pour répondre aux impératifs d'urgence. Par ailleurs, considérant que la rédaction retenue posait des difficultés opérationnelles, notamment au regard

avant la décision de toute interdiction. Enfin, le Sénat a adopté un amendement ayant un lien avec l'interdiction des néonicotinoïdes réaffirmée dans ce texte. Le principe d'une interdiction d'un produit phytopharmaceutique en raison de ses dangers pour l'environnement ou pour la santé ne doit pas pénaliser uniquement les agriculteurs français. Nous avons donc adopté à l'unanimité un amendement essentiel rappelant explicitement au ministre de l'agriculture, si besoin en était, qu'il dispose du pouvoir, en cas de danger sanitaire ou environnemental et en l'absence de mesure européenne, de suspendre les importations de denrées alimentaires ne respectant pas les normes européennes, notamment en raison de l'usage de produits phytopharmaceutiques interdits. C'est une avancée en matière de lutte contre les importations déloyales et un signal fort envoyé par la France à l'Union européenne,

qui devront respecter des délais imposés par l'urgence, les betteraviers et- j'y insiste -les industriels attendent l'annonce d'un plan d'indemnisation pour les dissuader de ne pas planter l'année prochaine. D'autres filières

mixte paritaire permet de faire du conseil de surveillance une instance de suivi de toutes les filières ayant utilisé dans le passé des néonicotinoïdes. Sur invitation de son président, cette instance pourra ainsi étudier les avancées de la recherche sur les autres filières, comme la filière de la noisette, sans pour autant leur octroyer de dérogations. Ainsi les plus petites filières, moins puissantes mais tout aussi importantes pour la diversité de l'agriculture et la régionalisation de celle-ci, pourront-elles être entendues et suivies. Enfin, vous le savez, monsieur le ministre, nous avons longuement insisté sur une véritable stratégie de recherche

venir. Pour aujourd'hui, il me semble que le texte issu de la commission mixte paritaire sur ce projet de loi est équilibré. Il apporte une réponse pragmatique et adaptée à la crise connue par la filière betteravière,

ministère de l'agriculture et de l'alimentation,

d'un engagement résolu en faveur de la transition agroécologique et d'une agriculture moins dépendante de l'ensemble des intrants.

être plus précis, ce projet de loi réintroduit, comme c'est déjà le cas pour de nombreux États membres, et jusqu'en 2023 au maximum, la possibilité de recourir au fameux article 53 du règlement européen et de solliciter des dérogations

votre attention sur le fait qu'il s'insère dans un plan global, qui comprend notamment 7 millions d'euros supplémentaires mobilisés au travers d'un programme de recherche publique et privée visant à accélérer l'identification d'alternatives véritablement efficaces et leur déploiement en conditions réelles. Ce plan comprend également des engagements pris par la filière au travers d'un plan d'action et de prévention. Le suivi de ces engagements, que ce soit sur le volet de la recherche ou sur celui du plan de prévention prévu par la filière,

Le projet de loi a fait l'objet de nombreux échanges tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez adopté la semaine dernière trois évolutions améliorant grandement le caractère opérationnel du futur Je pense à l'élargissement du conseil de surveillance, à l'encadrement du délai dans lequel il doit rendre son avis et à l'avancée de l'entrée en vigueur de la loi au 15 décembre

visant à clarifier encore davantage la mise en oeuvre de la future loi. Je souscris aux précisions apportées à la composition du conseil de surveillance : elles permettront notamment une nomination de ses membres explicitée et sécurisée. Je prends également acte de l'ajout d'un article rappelant la faculté pour le ministre de l'agriculture, mais aussi pour son collègue de la consommation, de prendre des mesures conservatoires afin de suspendre l'introduction, l'importation et la mise en marché en France de denrées

probablement jamais dans le futur -de pays fort et de civilisation forte sans une agriculture forte. Bravo ! Pour que notre pays soit fort, nous avons besoin d'une agriculture forte, permise par ces femmes et ces hommes qui,

encore une fois, un manque criant de moyens pour le développement de l'agriculture biologique et de l'agroécologie, en particulier dans le domaine de la recherche.

Il ne s'agit pas non plus d'une porte ouverte vers davantage de dérogations, puisque le texte les circonscrit aux seules betteraves sucrières. Il précise, en outre, clairement que les dérogations d'utilisation de produits phytopharmaceutiques ne seront possibles que sur décision commune des ministères de l'agriculture et de la transition écologique. Le comité d'évaluation des avancées de la filière aura un rôle essentiel : la dérogation sera circonscrite à la seule betterave sucrière et limitée dans le temps, jusqu'en 2023. Seul l'enrobage des semences sera possible, à l'exclusion de toute pulvérisation. Les semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d'insectes pollinisateurs seront temporairement interdits après l'emploi de ces semences. Ces derniers jours, nous avons entendu des propos qui minimisaient l'impact de la jaunisse sur les cultures betteravières et traitaient avec légèreté la perte des exploitants. Pourtant, au moment où le pays se reconfine, la préservation de nos richesses et champions nationaux est d'autant Au 20 octobre dernier, par exemple, selon les chiffres issus des délégués interministériels de la filière betterave-sucre-alcool, certaines pertes pouvaient atteindre de 70 % à 80

habilitant le pouvoir exécutif à suspendre ou à fixer les conditions particulières à l'introduction, l'importation et la mise sur le marché, en France, de denrées alimentaires ou de produits agricoles qui contiennent des substances interdites sur notre sol.

Cette garantie est essentielle pour les agriculteurs : il faut harmoniser les normes de production à l'échelle européenne. Le récent accord que vous avez obtenu dans la négociation de la politique agricole commune, s'inscrit tout à fait dans cette exigence,

À terme, personne ne l'ignore, les betteraviers ne pourront pas tenir face à une compétitivité agressive et à une production de plus en plus intensive et à bas coût. Si nous avions eu ce débat de fond, nous aurions pu coconstruire des propositions pour pérenniser la filière.

L'Allemagne a, elle, dès le départ, privilégié la lutte ciblée par pulvérisation. Je vous entends, monsieur le ministre, et je ne doute pas de votre volonté de faire au mieux, mais je crois que vous vous trompez.

la commission mixte paritaire est parvenue à un accord. Même si le Parlement doit faire face à une actualité chargée, entre l'urgence sanitaire et les exigences du calendrier budgétaire, ce texte ne doit pas pour autant être traité avec légèreté. Avant de l'adopter, nous devons mesurer l'étendue de la brèche qu'il ouvre dans notre législation. De très nombreux acteurs agricoles et économiques ont, malgré leurs réticences, appliqué l'interdiction des néonicotinoïdes. Ils se sont saisis des quatre années de transition pour revoir leurs pratiques et rechercher des alternatives. Quel message leur envoyons-nous : qu'en s'abstenant de tels efforts, ils auraient pu obtenir de pouvoir déroger à la loi ? Plus largement, un tel retour en arrière est un précédent redoutable pour toutes nos prochaines législations environnementales. Avec ce projet de loi, le Gouvernement ne tourne pas seulement le dos au long processus qui a conduit à la loi de 2016 sur la biodiversité, il enterre aussi un principe fort, inscrit depuis 2005 dans notre loi fondamentale, au sein de la Charte de l'environnement : « Les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. »

nier les « besoins du présent » auxquels ce texte prétend répondre. Il convient d'aider, sans délai, une filière qui craint une baisse de 15 % de son volume de production en 2020, en raison de la crise de la jaunisse de la betterave. Pour autant, la réponse à ce besoin immédiat ne peut évidemment pas être l'utilisation de produits qui n'auront d'effet que sur la prochaine récolte.

Les premières fermetures d'usine et suppressions d'emploi ont eu lieu alors que les néonicotinoïdes étaient encore utilisés par les betteraviers. Comment croire alors que leur réintroduction sera une réponse à des difficultés d'ordre structurel ? Selon nous, une réponse à la hauteur des enjeux consisterait plutôt à accompagner la filière vers une montée en gamme de la production sucrière, une véritable structuration et la mise en oeuvre de pratiques agriculturales adaptées pour faire face aux ravageurs. Ainsi, même au prix d'une régression environnementale qui fera précédent, ce projet de loi ne répond ni aux besoins immédiats ni aux besoins profonds de la filière betterave-sucre. La Constitution prévoit que « la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation

Ce projet de loi est une défaite magistrale ; c'est une défaite sanitaire et environnementale. Ainsi, nous n'honorerons pas la promesse faite en 2016 de commencer à réparer le monde, à changer les pratiques agricoles en abandonnant les insecticides systémiques et en explorant d'autres voies, voies, l'agroécologie par exemple, celles qui parient sur la diversité du vivant, en laissant opérer les petits artisans minuscules que la nature nous offre dans les écosystèmes, où tout est en interaction et en interdépendance

en matière de droit de l'environnement. Une « écologie de l'action et du réel », c'est un changement ambitieux des pratiques, qui ne s'affranchit pas des recommandations sanitaires et qui sait écouter : écouter la nature, écouter les véritables besoins des agriculteurs, mais aussi écouter la communauté scientifique, qui est, sur ce point, unanime. Le danger des semences enrobées de néonicotinoïdes est établi, avéré. Une étude récente de chercheurs du CNRS montre que l'imidaclopride est un produit toxique qui se diffuse largement hors des parcelles traitées. C'est un constat grave. Ces néonicotinoïdes se retrouvent à des taux très élevés, notamment dans les vers de terre, pourtant artisans essentiels de nos écosystèmes. On imagine facilement les effets délétères non seulement pour ces organismes, mais encore pour leurs prédateurs occasionnels que sont les oiseaux. vous apprêtez ainsi à acter la contamination généralisée des sols, censés être exempts de substances de synthèse. Sous les assauts répétés et corrosifs des néonicotinoïdes, les sols ne sont tout simplement plus vivants.

s'inquiètent du peu de cas que nous, les politiques, faisons de ce qu'ils nous disent, notamment sur les impacts que peuvent avoir nos décisions sur la santé humaine. Si nous n'avons pas le monopole de l'écologie, vous n'avez pas le don de la clairvoyance. Voter ce texte, c'est participer au déclin écologique et à une certaine forme de résignation économique. Vous faites le choix d'une solution court-termiste et de facilité. Nous n'entérinerons pas la réintroduction d'un poison dans le sol, pour la simple et bonne raison qu'il est une menace pour la chaîne du vivant. Je finirai en citant Jean-Marie Pelt et Gilles-Éric Séralini qui disent, à propos de l'édifice compliqué du vivant : « nous sommes en train d'[ ...] ôter les briques les unes après les autres en ignorant les conséquences de ce démontage à l'aveuglette, qui brise un à un les liens unissant la chaîne des êtres vivants. » La discussion

Décidément, la défense de la biodiversité et la santé des agriculteurs et des consommateurs ne font pas le poids face à quelques tonnes de betteraves à l'hectare. C'est une reculade lourde de sens et de conséquences Mes chers collègues, nous vous aurons alertés. La boîte à dérogations est ouverte. Demain, grâce à l'agriculture hyperconnectée, vous enverrez vos drones polliniser les cerisiers, Il s'agit d'une nouvelle illustration de vos choix politiques : vous êtes parfaitement conscient de la nocivité du produit, mais vous le réintroduisez malgré tout. Pourquoi ? Pour conforter la filière française dans une course sans fin à la compétitivité ? Pour privilégier le rendement maximal et le court terme ?

Le scrutin est clos. J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée

sur la proposition de loi relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ». Cet accord, qui est le fruit d'échanges nourris avec notre collègue députée Marie-Christine Verdier-Jouclas, auteure et rapporteure du texte pour l'Assemblée nationale, et avec le Gouvernement, devrait nous conduire à adopter, une dernière fois en ce qui nous concerne, cette proposition de loi. Malgré l'effet de loupe médiatique qui a fait porter l'essentiel des débats sur son titre II, relatif à la prolongation et à l'extension de l'expérimentation « zéro chômeur de longue durée

Le Sénat s'était opposé à ce que la participation des départements au financement de l'expérimentation soit obligatoire et fixée par décret. Ce point s'est révélé la divergence la plus difficile à surmonter, l'Assemblée nationale souhaitant laisser au Gouvernement la possibilité d'imposer par décret le montant de la participation exigée des départements. De notre côté, il ne nous avait pas paru acceptable que les départements puissent être tenus de participer financièrement, à hauteur d'un montant encore inconnu, à une expérimentation créée par l'État et résultant de la volonté de territoires. Le compromis auquel nous sommes parvenus consiste à accepter que la participation financière des départements soit déterminée par décret, mais à faire de l'accord du président du conseil départemental un prérequis pour qu'un territoire soit candidat à l'expérimentation. Sur proposition de l'Assemblée nationale, nous avons plafonné le montant maximal que le décret pourra imposer. Ce plafond est particulièrement élevé, puisqu'il s'établit au niveau du revenu de solidarité active (RSA) pour chaque personne embauchée, qu'elle ait précédemment été allocataire du RSA ou non. Il n'apparaît donc pas à mes yeux comme une garantie et il reviendra Il n'apparaît donc pas à mes yeux comme une garantie et il reviendra à chaque département d'apprécier si la participation à cette expérimentation est cohérente avec sa politique en matière d'insertion.

de trente nouveaux territoires constituait un maximum. J'espère que, si le nombre de soixante territoires expérimentateurs est un jour atteint, les demandes de dérogation qui pourront être adressées au Gouvernement seront examinées avec rigueur s'agissant du respect du principe de non-concurrence entre les entreprises à but d'emploi (EBE) et les entreprises locales, notamment celles de l'économie sociale et solidaire, et que le travail d'évaluation continuera à se poursuivre avec attention et objectivité.

Ainsi, le texte prévoit la possibilité, rétablie par le Sénat, de déroger, à titre exceptionnel, pour les salariés seniors rencontrant des difficultés particulières, à la durée maximale de vingt-quatre mois de renouvellement des CDD au-delà de l'âge de 57 ans, en complément de la faculté de conclure un « CDI inclusion senior », dans les entreprises d'insertion, les ateliers et chantiers d'insertion et les associations intermédiaires. Sur ce point de divergence, nos discussions avec l'Assemblée nationale nous ont permis de rapprocher nos points de vue. Les précisions apportées à la procédure du « Pass IAE », à l'article 1, figurent à l'identique dans le texte de la commission mixte paritaire, comme l'équilibre trouvé par le Sénat à l'article 2 concernant la possibilité pour le préfet d'accorder des dérogations au plafond de 480 heures de mise à disposition applicable aux associations intermédiaires. À l'article 3, le texte reprend les garde-fous apportés par le Sénat au cadre de l'expérimentation du « contrat passerelle », qui n'était pas accueillie favorablement par les réseaux de l'IAE. Nous avons introduit une condition d'ancienneté de quatre mois dans un parcours d'IAE pour les bénéficiaires, limité la durée de la mise à disposition à trois mois renouvelables et prévu de dispenser de période d'essai le salarié en cas d'embauche par l'entreprise utilisatrice, ce qui semble avoir rassuré les acteurs.

entre un contrat d'insertion et un CDI ou un CDD à temps partiel. Ce dispositif a également été retenu par la commission mixte paritaire. L'ensemble de ces mesures doit être envisagé en lien avec l'effort financier important consenti en faveur de l'IAE dans le cadre du plan de relance et de la « stratégie pauvreté » et devrait contribuer à soutenir les initiatives de terrain et à ouvrir le champ des possibles dans ce secteur. Nous saluons ces avancées, notamment sur le plan budgétaire. J'en viens au titre III et à l'article 7, relatif à l'articulation avec les allégements généraux de cotisations sociales du « bonus-malus » de contributions d'assurance chômage portant sur les contrats courts. Je rappelle que la commission des affaires sociales avait supprimé cet article afin de réaffirmer son opposition au bonus-malus et de tenir compte de la concertation en cours sur la réforme de l'assurance chômage. Ce dispositif étant déjà inscrit dans le droit et étant prêt pour une entrée en vigueur au début de l'année 2021, il a cependant paru préférable de rétablir l'ajustement proposé, faute de quoi l'application du bonus-malus serait préjudiciable aux entreprises, notamment les plus vertueuses. Cet article prévoit également d'exonérer les contrats d'insertion du bonus-malus, ce qui semble raisonnable. Il est entendu que cela ne vaut pas approbation du principe du bonus-malus et je demeure convaincue, sur le fond, que ce n'est pas la solution appropriée pour lutter contre les abus du recours aux contrats courts. l'article 9, l'expérimentation d'un contrat de professionnalisation « sur mesure », créée par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sera bien prolongée de deux ans, comme l'a proposé le Sénat, pour permettre son appropriation par les SIAE. Enfin, à l'article 9 , le Sénat avait introduit, sur l'initiative du Gouvernement, une expérience visant, en complément des initiatives existant déjà dans certaines branches, à encourager le dialogue social au sein des SIAE et à permettre une meilleure représentation des salariés en parcours d'insertion. a retenu une nouvelle rédaction de cet article, qui tend à prévoir, au lieu d'une instance de dialogue social, la création d'une commission « insertion » au sein du comité social et économique (CSE), ce qui répond davantage aux attentes des partenaires sociaux. Ce dispositif aura l'avantage d'être moins lourd pour l'employeur, tout en remplissant les mêmes objectifs.

en préambule, permettez-moi d'exprimer à la représentation nationale la solidarité du Gouvernement dans cette nouvelle phase de confinement. Comme l'a dit le Premier ministre, nous devons redoubler d'attention pour les publics les plus fragiles et les plus éloignés de l'emploi. Pour eux, la solidarité nationale doit continuer à se déployer pleinement. Je pense tout d'abord aux jeunes, mais aussi aux demandeurs d'emploi de longue durée et aux personnes fragiles. Dans ce nouveau contexte, les deux dispositifs renforcés par cette proposition de loi trouvent plus que jamais leur utilité. Tout au long du processus parlementaire, un travail constructif a été mené par les députés et les sénateurs de tous les groupes : chacun a pu apporter sa pierre à l'édifice d'ensemble.

je profite de l'occasion pour vous souhaiter un très bel anniversaire. Je note que le texte de la commission mixte paritaire reprend l'ensemble des apports du Sénat. À son tour, la commission mixte paritaire a travaillé à l'équilibre définitif du texte, pour aboutir à une version qui respecte à la fois le « pacte d'ambition pour l'IAE » et l'esprit des fondateurs de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ». Les deux chambres ont su aboutir à un texte pragmatique, nécessaire, utile, émanant des acteurs de terrain. Je remercie donc la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 28 octobre dernier d'être parvenue à cet accord. Nous avons abouti à un texte adapté aux circonstances. Aujourd'hui, son adoption finale est dans l'intérêt de tous et de tous les territoires. Ce texte est, en effet, un bel objet en faveur de l'emploi pour tous et de l'égalité des chances. Vous le savez, il renforce deux très beaux outils, qui appliquent des méthodes complémentaires pour insérer dans l'emploi les personnes qui en sont les plus éloignées. Le titre I est consacré au renforcement du secteur de l'insertion par l'activité économique. Les structures d'insertion par l'activité économique vont ainsi voir leurs règles de recrutement simplifiées, grâce à la suppression de l'agrément préalable délivré par Pôle emploi, ce qui leur permettra d'embaucher plus rapidement. Le titre II a pour objet de prolonger et d'étendre l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée Cette expérimentation se déploiera désormais dans soixante territoires, cinquante nouveaux venant s'ajouter aux dix premiers, qui sont reconduits. Je salue le travail et la persévérance de Laurent Grandguillaume, président de l'association Territoires zéro chômeur

Pour chacun des trois titres de cette proposition de loi, la commission mixte paritaire a su apporter des avancées majeures. Au titre I, consacré à l'insertion par l'activité économique, le texte issu de la maintient le « CDI inclusion » destiné aux seniors, lequel apporte une sécurisation du travail de ces personnes jusqu'à leur retraite. Tout salarié d'une structure d'insertion par l'activité économique âgé de plus de 57 ans au moment du renouvellement de son parcours pourra se voir proposer un CDI, si sa situation ne lui permet pas de retrouver un emploi dans le secteur de droit commun. Conformément à la volonté du Sénat, ce nouveau contrat coexistera avec les contrats à durée déterminée insertion, qu'il est possible de renouveler par dérogation à partir de 50 ans. encore, députés et sénateurs ont également su s'accorder pour doser l'encadrement de l'expérimentation du « contrat passerelle ». L'objectif est de permettre une transition progressive entre un contrat d'insertion et un CDI ou un CDD à temps partiel. Sur ce sujet, nous saluons le travail d'écoute de Mme le rapporteur, qui a su aménager le « contrat passerelle » et introduire un dispositif complémentaire de « temps cumulé », afin de laisser aux acteurs le libre choix des outils. Concernant le titre II et l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », la commission mixte paritaire a permis plusieurs apports décisifs. Premièrement, la commission mixte paritaire a rétabli le caractère obligatoire du financement des départements, en revenant au texte de l'Assemblée nationale, mais en ajoutant deux points la fixation par décret du niveau de cette participation et le plafonnement de celle-ci. Nous entendons, bien sûr, les inquiétudes sur le niveau de dépenses que devront supporter les départements, raison pour laquelle nous travaillerons avec l'Assemblée des départements de France à la meilleure rédaction possible du décret. Deuxièmement, la commission mixte paritaire précise que l'accord du président du conseil départemental est requis pour qu'un territoire se porte candidat à l'expérimentation. Nous saluons l'accord et l'équilibre trouvés. Ils ont d'ailleurs été salués par l'association Territoires zéro chômeur de longue durée elle-même. Cette solution préserve à la fois l'esprit même du texte et la compétence des départements en tant que chefs de file de la politique d'insertion dans les territoires. D'une part, nul ne pourra imposer aux départements de participer financièrement à une expérimentation qui serait incohérente avec la politique qu'ils définissent librement en matière d'insertion. D'autre part, conformément à leur compétence en matière d'insertion, il est cohérent que les départements participent au financement des expérimentations qui ont lieu sur leur territoire. Respect de la compétence des départements et engagement de tous les acteurs de l'insertion dans les projets territoriaux : c'est tout l'équilibre qui a été trouvé en commission mixte

Conjointement avec le Gouvernement, la commission mixte paritaire est finalement parvenue à trouver une solution juridiquement satisfaisante, en permettant d'élargir le nombre de territoires au-delà de soixante si cela était nécessaire, et de l'insertion, Élisabeth Borne, s'y était fermement engagée à l'Assemblée nationale. Au titre III a été introduite une avancée majeure pour l'insertion par l'activité économique, à travers la mise en place d'un dialogue social pour les salariés en insertion, sous la forme d'une expérimentation de trois ans. Les structures d'insertion par l'activité économique pourront mettre en place, au sein du CSE, une commission « insertion », qui débattra des conditions de travail des salariés en insertion et de la qualité des parcours proposés par les structures. Les salariés en insertion pourront, enfin, prendre part à un véritable dialogue social, avec tous les intérêts que comporte un engagement syndical en termes de reconnaissance et d'émancipation pour la suite de leur parcours professionnel. Je salue ici l'engagement de Mme le rapporteur Frédérique Puissat, qui a soutenu cette expérimentation lors des discussions en séance publique au Sénat, puis en a amélioré le contenu lors Ce texte prouve la volonté du Gouvernement d'agir en faveur de l'emploi pour tous. Il s'inscrit dans une ambition plus large, visant à développer des solutions d'insertion dans l'emploi pour les personnes plus fragiles. Dans le cadre de « France Relance » est prévue la priorisation de 35 000 places dans l'insertion par l'activité économique au bénéfice des jeunes. En outre, conformément aux annonces récentes du Premier ministre sur les mesures de prévention et de et de lutte contre la bascule dans la pauvreté, en date du 24 octobre dernier, est également prévue l'ouverture de 30 000 places supplémentaires dans l'IAE. Cette volonté politique sans précédent en faveur de l'insertion par l'activité économique est parfaitement complémentaire de cette proposition de loi. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez l'opportunité de voter des outils concrets et adaptés aux circonstances de la crise que traverse la France. Nous nous attacherons à prendre les textes d'application nécessaires. Au nom du Gouvernement, je renouvelle nos remerciements à l'ensemble des parlementaires et à Mme le rapporteur pour leur travail d'enrichissement du texte. Mesdames, messieurs les sénateurs, afin d'oeuvrer à ce que la relance de notre économie soit la plus inclusive possible, je vous demande une adoption définitive de cette proposition de loi la plus large possible. Très bien

Je reprends ces mots du président du Conseil de l'inclusion dans l'emploi pour introduire mon propos, car j'ai le sentiment qu'ils reflètent parfaitement l'esprit de cette proposition de loi et de l'accord que nous avons trouvé en commission mixte paritaire. Alors que 4,2 millions de personnes se trouvent éloignées de l'emploi, dont 2,7 millions depuis plus d'un an, la proposition de loi vient apporter une réponse concrète, ambitieuse et innovante dans la lutte contre le chômage de longue durée, véritable fléau de notre société. Elle s'inscrit dans la logique du plan de relance et dans la volonté du Président de la République d'intégrer 140 000 personnes supplémentaires dans les parcours d'insertion et les entreprises adaptées. Elle vient aussi compléter le dispositif de 300 millions d'euros en faveur des structures d'insertion que vous avez annoncé, madame la ministre. L'insertion par l'activité économique constitue, en effet, une riposte efficace, qui concilie à la fois l'économie, le social et le territorial. Nous saluons le compromis trouvé, qui préserve l'esprit même du texte en réintégrant notamment l'obligation de financement des départements concernés par l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » et l'absence du préfet dans son copilotage, démontrant ainsi la confiance que nous souhaitons donner aux territoires et aux acteurs locaux. La lutte contre le chômage de longue durée nécessite de faire preuve de créativité et d'innovation, en s'appuyant sur les territoires et en associant l'ensemble des acteurs : je pense aux entreprises, aux associations et aux collectivités territoriales. Grâce à ce compromis, nous concrétisons des avancées notables pour lutter contre l'isolement des personnes privées d'emploi en instaurant le « CDI inclusion senior » à destination des personnes de plus de 57 ans. Au moment où le marché de l'emploi est durement frappé par la crise sanitaire, il est nécessaire de renforcer les dispositifs existants pour favoriser le retour à l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées. Je pense, bien sûr, aux chômeurs de longue durée, mais aussi aux bénéficiaires des minima sociaux, aux personnes en situation de handicap et aux parents isolés. Les dispositions de cette proposition de loi, telles que l'extension de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » à cinquante nouveaux territoires, le développement des structures d'insertion par l'activité économique, grâce à la suppression de l'agrément préalable délivré par Pôle emploi, et l'expérimentation du « contrat passerelle », constituent des réponses fortes dans la lutte contre le chômage de longue durée. Par ailleurs, en permettant à de nouveaux territoires qui souhaitent bénéficier de l'expérimentation d'être habilités par décret, la clause de revoyure constitue, à nos yeux, une avancée notable.

Enfin, nous nous réjouissons de voir aboutir cette proposition de loi et saluons le travail des rapporteurs en vue de la recherche d'un compromis ambitieux. Nous formons le voeu que cette expérimentation puisse être généralisée sur le long terme, afin de permettre une meilleure insertion à ceux qui demeurent éloignés de l'emploi, grâce au travail des associations, des collectivités et de tous les acteurs de terrain mobilisés. La parole

la crise sanitaire que nous connaissons depuis le printemps dernier s'accompagne d'une crise économique et sociale chaque jour plus prégnante. Selon les associations caritatives, cette crise a fait basculer dans la pauvreté 1 million de Français, qui rejoignent ainsi les 9,3 millions de personnes vivant déjà au-dessous du seuil de pauvreté. Le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire augmente dramatiquement : au mois de septembre dernier, ils étaient 8 millions, contre seulement- si j'ose dire -5,5 millions en 2019. Dans ce contexte, s'il est un sujet qui doit faire consensus, c'est bien la lutte contre le chômage ! Notre groupe est convaincu que ce texte apportera les outils nécessaires pour aider les personnes les plus éloignées du monde du travail à retrouver un emploi. C'est pourquoi nous nous félicitons de ce que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord et nous saluons le compromis ainsi trouvé. Nous approuvons notamment le maintien du dispositif de « temps cumulé », qui facilitera la transition de l'insertion par l'activité économique vers le secteur marchand. Nous accueillons également très favorablement la mise en place d'une expérimentation visant à encourager le dialogue social au sein des structures d'insertion par l'activité économique. Nous nous félicitons surtout de ce que la commission mixte paritaire ait ouvert la voie à une augmentation dérogatoire par décret du nombre de territoires concernés par l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée ». Nous étions très nombreux, dans cet hémicycle, à le réclamer. Nous pensons, en effet, qu'aucun territoire remplissant les conditions pour en bénéficier ne doit être laissé sur le bord du chemin. Certes, plusieurs études ont pointé du doigt le coût de ce dispositif, mais, comme je l'ai rappelé en première lecture, celui-ci ne doit pas seulement se résumer à son aspect financier. En permettant à des personnes particulièrement éloignées du monde du travail de retrouver un emploi, cette expérimentation leur permet aussi et surtout de retrouver leur dignité, de reprendre confiance en elles. N'oublions pas que ces personnes sont très souvent « cassées » par des années de chômage, des carrières brisées, des fractures de vie. En adoptant cette proposition de loi, nous réunissons les conditions nécessaires à la réussite de cette expérimentation, qui repose sur l'implication de chacun et les compétences de tous. Cette seconde phase va pouvoir s'appuyer sur les dix territoires déjà engagés, qui ont eu un véritable rôle de laboratoires, mettant en lumière les améliorations à apporter apporter : locaux adaptés aux besoins, nécessité de mettre l'accent sur la formation ou encore renforcement des conditions d'habilitation des territoires pour ne laisser partir que les territoires prêts qui se sont donné les moyens de réussir. Les territoires qui postulent pour la seconde phase de l'expérimentation auront été préparés grâce à l'expérience qu'ils auront tirée de la première phase. Cette proposition de loi intervient dans une période où nous avons plus que jamais besoin d'ouvrir la porte à des méthodes novatrices. Certains qualifient toujours

Ce texte me tient à coeur et je suis heureuse de pouvoir prendre part à nos débats aujourd'hui. Dans mon territoire, particulièrement touché par la désindustrialisation, les acteurs de l'activité économique sont demandeurs de ce type d'expérimentation pour essayer d'agir sur les freins du retour à l'emploi.

Le Gouvernement a ajouté le renforcement du contrôle des chômeurs par les agents de Pôle emploi avec l'instrument des carnets de bord. Il a également transféré la responsabilité de la formation professionnelle aux salariés eux-mêmes, en leur demandant d'utiliser leurs crédits du compte personnel de formation avant toute demande de prise en charge financière par les régions ou Pôle emploi.

Votre « contrat passerelle » est un cache-misère des politiques qui ont supprimé les départs en retraite anticipée et des décotes imposées aux départs sans carrière complète. En réalité, vous allez affaiblir les plus fragiles, et particulièrement les femmes seniors, comme si nous ne connaissions pas une grave crise économique avec la covid-19 et comme si les 800 000 personnes supplémentaires au chômage n'allaient pas renforcer les rangs des 2 millions de femmes et d'hommes déjà éloignés de l'emploi avant la crise sanitaire ! Ces 2 millions de personnes éloignées de l'emploi, ce sont des chômeuses et des chômeurs de longue durée, mais également des gens en situation de handicap, des bénéficiaires des minimas sociaux ou encore des parents isolés. isolés. Nous ne sommes pas dupes : l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » ne résoudra pas la crise sociale rencontrée dans nos territoires. Ces initiatives locales servent à redonner de l'espérance à celles et ceux qui ont le sentiment que les services publics ont abandonné, publics ont abandonné, mais ne peuvent remplacer une politique publique de l'emploi à l'échelon national qui garantisse à chacun de pouvoir évoluer dans sa vie professionnelle selon ses aspirations, sans perte de revenu et sans jamais passer par la case « chômage La sécurité d'emploi et de formation permettrait de changer radicalement de logique. Dans le cadre d'un nouveau service public de l'emploi et de la formation, chaque personne ayant terminé sa scolarité pourrait alterner périodes de travail salarié et périodes de formation rémunérées, à la faveur d'une réduction générale du temps de travail permise par les gains de productivité qu'apportent les nouvelles technologies.

La parole est à Mme Élisabeth Doineau.

J'ai eu la chance de participer à la commission mixte paritaire qui a permis d'aboutir à ce texte commun. Dans la continuité de l'esprit de dialogue entre le terrain et la représentation nationale qui émane de cette proposition de loi, je me félicite que le Parlement se soit entendu sur une version partagée. Je tiens à saluer tout particulièrement Frédérique Puissat, notre rapporteur, pour son travail actif, mené de concert avec son homologue de l'Assemblée nationale. C'est un grand pas dans la lutte contre l'éloignement de l'emploi. L'extension de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » ouvre ainsi la possibilité de réaliser un travail sur mesure, au plus près du terrain, tout en posant des jalons nécessaires dans la refondation de la politique de l'emploi. Parmi les modifications notables apportées par la commission mixte paritaire figure la possibilité d'augmenter de manière dérogatoire, par décret, le nombre de territoires concernés par l'expérimentation. Dans l'attente du rapport final du comité scientifique, il s'agit de la solution la plus opportune et sans doute la plus sécurisante. La jauge de soixante territoires en expérimentation était vue comme injuste vis-à-vis des cent vingt candidats déjà déclarés. L'augmentation dérogatoire permettra de continuer de répondre aux besoins identifiés localement et partagés collectivement. Le texte prévoit que le montant de la participation financière des départements au financement des emplois créés dans le cadre de l'expérimentation puisse être puisse être fixé par un décret et fait de l'accord du président du conseil départemental une condition requise pour qu'un territoire se porte candidat. C'est un compromis qui peut nous satisfaire- je m'en contenterai donc-, le département conservant ainsi sa liberté d'apprécier si l'expérimentation est cohérente ou non avec sa politique d'insertion. Je veux rappeler que la loi du 1 décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion affirmait déjà le rôle de chef de file du conseil départemental en matière de politiques d'insertion. il peut signer- ce qu'il fait la plupart du temps -avec des partenaires institutionnels un pacte territorial d'insertion pour définir, animer et coordonner les politiques d'insertion du département. C'est un véritable outil d'insertion coconstruit avec une pluralité d'acteurs autour d'un projet commun qui a fait ses preuves. Selon moi, ce pacte territorial d'insertion peut inclure une démarche « territoires zéro chômeur de longue durée Ainsi n'était-il pas opportun d'apporter par la loi des obligations supplémentaires aux collectivités territoriales. En tant que représentants des territoires, c'est à nous de leur faire confiance. Aussi, je me réjouis que le Parlement ait su respecter cet équilibre. concerne le détail des articles, il me semble que le Sénat, par la voix de son rapporteur, a apporté des améliorations visant à répondre aux interrogations des acteurs de terrain. Au sein du titre I, les mesures du Sénat visant à assouplir les dispositifs d'insertion par l'activité économique pour les salariés âgés de plus de 57 ans ou à permettre de cumuler contrat de travail de droit commun et contrat d'insertion ont été conservées. À l'article 3 , le cadre de l'expérimentation du « contrat passerelle » a notamment été précisé pour répondre aux nombreuses oppositions émanant des réseaux de l'IAE. En complément de ce contrat, la Haute Assemblée a introduit un dispositif de « temps cumulé » afin de permettre une transition progressive entre contrat d'insertion et CDI ou CDD à temps partiel. Ce dispositif facilitera le rapprochement entre l'IAE et le secteur marchand. Enfin, le Sénat a introduit, à l'article 9, une expérimentation visant à encourager le dialogue social au sein des structures de l'IAE et à permettre la représentation des salariés en parcours d'insertion. Ainsi est créée une commission « insertion » au sein du comité social et économique (CSE), plutôt qu'une instance de dialogue social. Opposé au bonus-malus, le Sénat a supprimé l'article 7 relatif à l'articulation avec les allégements généraux généraux de cotisations sociales du bonus-malus de contributions d'assurance chômage portant sur des contrats courts. Pour aboutir à ce texte de compromis, la commission mixte paritaire a réintroduit l'article. L'ajustement proposé vise à ne pas pénaliser les entreprises, notamment les plus vertueuses. Pour conclure, face aux conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire, cette proposition de loi est une bouffée d'espoir. En mettant en oeuvre certaines mesures du pacte d'ambition pour l'insertion par l'activité économique et le deuxième volet de l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », elle participe à améliorer notre politique de l'emploi, notamment vers les personnes les plus fragiles.

cet hémicycle et en commission mixte paritaire à l'occasion de l'examen de la proposition de loi sur le renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée

L'adoption de ce texte nous paraît opportune et nécessaire. Nous nous sommes abstenus en première lecture, car nous étions en désaccord avec certaines des propositions de Mme la rapporteure. Cependant, des avancées notables sont intervenues dans le cadre de la commission mixte paritaire

Ces avancées concernent notamment la confiance renouvelée aux acteurs de l'insertion par l'activité économique au sein du dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée », la mise en place d'une clause de revoyure et l'instauration d'un financement par les départements sous certaines conditions,

Ainsi, pour ce qui est du nombre de territoires participant à cette expérimentation, la clause de revoyure permettra de ne pas laisser au bord du chemin les territoires investis dans la démarche d'intégration au sein de l'expérimentation. Nous sommes également satisfaits que la question du concours financier des départements- sous certaines conditions -ait été tranchée positivement. Nous avons cependant quelques regrets, notamment l'absence de financement des comités locaux pour l'emploi par le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée. La question des moyens alloués à ces comités locaux pour l'emploi était pourtant essentielle ils sont la véritable pierre angulaire de la dynamique territoriale que génère le projet. Il aurait fallu prévoir les moyens nécessaires à la bonne conduite de leurs missions et permettre au fonds d'expérimentation de financer une partie, et seulement une partie, de leurs charges de personnel. Nous pensons

Ces réserves ne nous empêchent pas de saluer l'adoption à venir de ce texte dont les enjeux sont plus que jamais d'actualité. Avec les difficultés qui se profilent pour des millions de Français dans le sillage de la crise sanitaire, nous avons plus que jamais besoin que se déploient les solutions innovantes de l'économie sociale et solidaire,

reculer de deux demain. L'année dernière, dans cette même enceinte, emmené par Joël Bigot, notre groupe a bataillé, avec d'autres, dans le cadre de l'examen du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, pour la création d'un fonds spécifique pour le réemploi solidaire.

Par ailleurs, je ne peux m'empêcher de remarquer, avec un peu de malice, que les contrats aidés sont rentrés dans les bonnes grâces du Gouvernement, alors qu'on ne leur trouvait plus aucune vertu en 2017.

Si nous saluons les avancées de la présente proposition de loi, nous nous devons aussi d'en appeler au Gouvernement pour qu'il garde à l'esprit la nécessité de maintenir un souci de cohérence dans le cadre des politiques qu'il choisit de mettre en oeuvre.

alors que la crise sanitaire fait basculer nombre de Français dans la précarité, il est plus que jamais urgent de trouver des solutions qui permettent de favoriser l'inclusion dans l'emploi et ainsi aider les populations fragilisées à retrouver leur autonomie et leur dignité par le travail. La proposition de loi déposée par notre collègue députée Marie-Christine Verdier-Jouclas constitue une réponse intéressante, qui contribuera à enrichir les dispositifs en direction des personnes les plus éloignées de l'emploi à travers deux leviers part, l'insertion par l'activité économique, d'autre part, l'expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée », dont la prolongation est sans nul doute une décision dont nous devons nous féliciter. En effet, cette initiative issue de la société civile permet de fournir un emploi durable à tous les demandeurs d'emploi qui en feraient la demande. La contribution financière des départements à ce dispositif constituait un sujet de désaccord entre les deux assemblées. La solution retenue, solution de compromis, est une obligation de participation financière associée à un accord préalable du département pour qu'un territoire puisse se porter candidat. Il sera également possible d'augmenter le nombre de territoires concernés par l'expérimentation, ce qui est aussi une bonne chose. En effet, seuls dix territoires étaient concernés par le premier volet de l'expérimentation. Le texte adopté prévoit d'accroître à soixante le nombre de territoires

En ce qui concerne le titre I consacré aux dispositifs d'insertion par l'activité économique, nous nous félicitons que les contributions du Sénat aient été reprises. Le dispositif de temps cumulé permettra de sécuriser la transition entre un contrat d'insertion et un emploi classique. Comme je l'ai indiqué lors de l'examen du texte en séance, ce dispositif se rapproche de celui qu'a proposé Claude Malhuret dans la proposition de loi qu'il a déposée le 13 octobre dernier et que je vous invite à cosigner, Il s'agit d'une demande d'expérimentation exprimée par les départements qui permettrait aux allocataires du RSA d'effectuer quinze heures de travail hebdomadaires pendant un an dans une entreprise, sans perdre le bénéfice du RSA, afin de sécuriser les démarches de retour à l'emploi et de les favoriser. Dans le contexte difficile que nous connaissons, toutes les initiatives comptent pour permettre aux personnes placées en situation de vulnérabilité économique de retrouver un revenu d'activité. Le 24 octobre dernier, le Premier ministre a annoncé les mesures de l'acte II du plan contre la pauvreté dans un contexte social particulièrement préoccupant. La crise sanitaire a fait basculer un million de Français dans la pauvreté, alors que la situation était déjà préoccupante, avec près de 15 % de nos concitoyens sous le seuil de pauvreté en 2018, selon l'Insee. La Banque de France confirme un taux de chômage supérieur à 10 % en 2020. Nous devons donc prendre la mesure de la situation et permettre à l'ensemble des acteurs de bonne volonté de se mobiliser sur le terrain, au plus près des besoins, pour lutter contre la précarité. Cette loi sera un très bon outil. Je salue tous les efforts

Il nous semble particulièrement important d'inclure dans l'emploi des chômeurs de longue durée non par des contrats précaires ou aidés, mais bien par des contrats à durée indéterminée, ce qui génère une dynamique très positive pour eux et, au-delà, pour leur territoire, pour tout l'écosystème local. Nous avions très fortement regretté que le Sénat ait sensiblement modifié le dispositif. Pour autant, le travail réalisé par la commission mixte paritaire nous satisfait. faut saluer la réintroduction du caractère obligatoire de la participation financière des départements à l'expérimentation. Nous avions fait des propositions pour qu'il soit préservé. Il en est de même de la suppression du copilotage des préfets avec les comités locaux,

permettent de mettre à disposition un salarié en insertion auprès d'entreprises de droit commun en vue de leur éventuelle embauche. Nous avions défendu la suppression de cette disposition, en accord avec les professionnels du secteur de l'insertion. Le dispositif proposé ne nous convient pas en ce qu'il ne remplit pas l'objectif de sécurisation des parcours et qu'il ne permettra pas de sortir les personnes concernées de la précarité. Toutefois,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de l'examen de cette proposition de loi, à la suite Je tiens tout d'abord à saluer le travail de notre rapporteur, Frédérique Puissat, qui s'est fortement engagée dans l'examen de ce texte. Elle a su trouver une position équilibrée qui a retenu l'approbation du groupe Les Républicains. Lors de nos débats, j'ai pu témoigner de la réussite du dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée », cette expérimentation étant menée dans un département dont je suis l'élu, les Deux-Sèvres.

Au-delà de ce cas particulier, il nous appartenait, en tant que parlementaires, de tirer les enseignements de presque cinq années de mise en oeuvre du dispositif, l'objectif étant d'organiser, si les retours étaient positifs, sa prolongation et son extension. Le Sénat s'est attaché à une étude objective des premiers éléments communiqués, sans s'arrêter à l'engouement suscité par le côté novateur de l'expérience. Il a ainsi analysé son efficacité sous deux aspects : le nombre d'emplois créés et le coût pour les pouvoirs publics. Cependant, l'essentiel n'est peut-être pas là. L'expérimentation, sans être le seul remède miracle au chômage de longue durée, a suscité une mobilisation collective dans des territoires parfois sinistrés économiquement et a permis de proposer un travail à des personnes en situation d'exclusion durable, avec toutes les conséquences financières et psychologiques que cela implique. Ces personnes ont retrouvé une place dans la société. Je peux en témoigner, notamment après suite de ce constat, le Sénat a décidé la prolongation de l'expérimentation en lui apportant plusieurs aménagements. Nous avons confié un rôle de suivi au fonds d'expérimentation qui remettra un rapport annuel retraçant le profil des personnes embauchées et les économies réalisées en termes de prestations sociales.

Nous répondons ainsi à une demande forte qui a donné lieu à de longs débats avec le Gouvernement. De nombreux territoires sont en attente : il ne faut pas briser cette dynamique. concerne le financement du dispositif, le Gouvernement souhaitait rendre obligatoire la participation des départements. En tant que représentant des territoires, le Sénat ne pouvait valider une telle proposition en l'état. Lors de l'examen du texte adopté en 2016, j'avais fait préciser que le dispositif serait principalement financé par l'État et que les collectivités territoriales pourraient participer, mais de manière volontaire. En effet, il ne peut être question d'imposer de nouvelles charges financières aux collectivités territoriales engagées dans le processus. La baisse des dotations de l'État et le surcroît de dépenses occasionné par la montée en charge des dépenses sociales ne laissent aucune marge de manoeuvre financière aux départements. Aussi la commission mixte paritaire a-t-elle proposé une solution de compromis : le département conserve son libre choix, mais, s'il accepte la candidature, il s'engage à participer au financement de l'expérimentation. En effet, comme l'a souligné notre rapporteur, on ne peut imposer au département de participer financièrement à une expérimentation qui ne serait pas cohérente avec la politique qu'il définit librement en matière d'insertion. Je tiens, à cet égard, à saluer les travaux et l'écoute de notre rapporteur qui lui ont permis de nous proposer des dispositions réellement adaptées aux réalités du terrain.

Le secteur de l'insertion par l'activité économique est en effet lourdement affecté par la crise sanitaire qui a provoqué la fermeture de nombreuses structures et la baisse de leurs résultats. Les mesures de simplification, les assouplissements et les nouveaux contrats prévus par la proposition de loi sont donc particulièrement bienvenus.

L'objectif est un retour durable à l'emploi, il me semble important de toujours le préciser. Le groupe Les Républicains va donc soutenir cette proposition de loi ainsi amendée.

emploi depuis plus d'un an. Il est avant tout urgent de relancer l'économie, de soutenir nos PME, nos TPE, nos artisans, nos commerçants, qui sont les véritables créateurs d'emplois, et ce dans le contexte de la crise sanitaire, qui perturbe profondément notre système économique. Ainsi précisée, la présente proposition de loi aura le soutien de notre groupe. En effet, si nous regrettons l'absence d'une réforme d'ampleur de la part du Gouvernement, nous approuvons toute initiative rassemblant les énergies au niveau local et destinée à permettre aux chômeurs connaissant le plus de difficultés de renouer avec une vie normale, c'est-à-dire une vie avec un emploi.

le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte.

tout particulièrement. C'est un texte important que vous venez d'adopter dans un contexte, hélas, de crise sanitaire et économique. Cette proposition de loi est un signe d'espoir et une réponse concrète pour les personnes éloignées de l'emploi, pour les personnes les plus fragiles. C'est un pas de plus pour ne laisser personne sur le bord du chemin, et je tiens à vous remercier pour son adoption très large. Mes chers

La séance est suspendue.